La séance est reprise. Mais, chers collègues, les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat, en l'absence d'observation, je considère ces conclusions comme adopté. L'ordre du jour appelle le débat sur les conclusions du rapport 5 plans pour reconstruire la souveraineté économique d'une demande de la commission des affaires économiques. Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire. De prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de 2 minutes l'orateur disposera alors à son tour du droit d'répartis pour une minute. Monsieur le Ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que ce Lucie aura retrouvé une place dans l'hémicycle. La parole et tout d'abord aux orateurs de la commission qui a demandé ce débat je passe la parole à Madame Hamel Gacquerre au nom de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, mes chers collègues, hier, le paracétamol les masques et les puces électroniques aujourd'hui la moutarde, l'huile de tournesol et le gaz, alors que les crises économiques, sanitaires, sécuritaires s'enchaînent, notre pays se redécouvre vulnérables comment avons-nous pu en arriver là et surtout de là des constats : comment sortir de cet état de dépendance qui nous coûte et nous contraint c'est ce sujet fondamental de souveraineté qui a occupé notre commission pendant près de 6 mois, le rapport présenté avec la présidente Sophie Primas une autre collègue Franck Montaugé nous a permis d'identifier précisément nos vulnérabilités dans différents secteurs et notre constat est alarmant car il révèle une perte d'autonomie transversales et profonde à l'heure où la guerre frappe aux frontières de l'Europe ou l'arme économique n'est plus taboue, les frontières entre économie réelle et économie numérique se brouille ou la valeur de l'énergie continue d'augmenter, où la concurrence internationale en matière de talent fait rage, il nous faut avoir le courage de regarder les choses en face, reconstruire notre souveraineté doit être avec la transition écologique, la priorité majeure de nos politiques publiques, c'est la raison pour laquelle notre commission a appelé à passer à l'acte du sursis au sursaut via 5 plan stratégique stratégique je souhaite évoquer ici 3 postulats sur lesquels reposent ces plans d'abord ne pas opposer les souverainetés, la France a besoin de l'Europe, pour être plus forte, il faut mobiliser ensemble avec nos voisins, davantage de moyens et d'innovation nombres de nos recommandations concernent l'action de l'Union européenne en matière de télécommunications de législations environnementales ou de projets industriels communs pour exemple 99 % du réseau Internet transite via les câbles sous-marins, contrôlé majoritairement par les Gafam pour les raisons pour des raisons évidentes de sécurité et de gestion des risques, il nous faut travailler à l'établissement d'un réseau indépendant de câbles sous-marins de télécommunications reliant entre les pays de l'Union européenne dans ce même registre, le transfert de données hors de France et de l'Union européenne ne cesse de croître, il faut rendre obligatoire la localisation, le stockage des données personnelles des citoyens et des entreprises européennes sur le sol de l'Union européenne, autre principe pour garantir notre souveraineté, une meilleure exploitation de nos forces et nos ressources, qu'elles soient minières humaine ou agricoles et ce dans le respect de l'environnement, plutôt que de choisir la dépendance aux importations et la politique pardon, qui en découle, vous le savez la France dépend à 100 % de la Chine pour les Terres rares et 80 % de l'Amérique du Sud pour le lithium intensif et par exemple le soutien au recyclage des métaux critiques et des biens industriels nous semble essentiel pour réduire notre dépendance : la question des compétences est également fondamentale, nous avons de fortes ambitions pour notre industrie, mais un employé sur 3 de l'industrie partira à la retraite d'ici 2030 et 50 % des métiers de l'industrie sont en tension, nous évoquons le développement de la filière nucléaire, mais avons-nous aujourd'hui les compétences suffisantes pour cela, il nous faut de matières urgentes repenser les filières et les diplômes de demain sur les métiers en tension, le numérique, la métallurgie, l'électronique pour finir dans le cadre de ce rapport, nous invitons à poursuivre l'effort de compétitivité d'ancrage de notre tissu économique, notre souveraineté ne repose pas que sur nos grandes entreprises françaises, même si elle joue un rôle moteur pour l'économie qu'il convient de les protéger, c'est aussi l'ensemble des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, les Start-Up innovantes, les exploitants agricoles qui garantissent au quotidien La résilience de notre économie et de notre société, il faut leur assurer un environnement compétitif dans lequel ils peuvent se développer sans craindre la justice fiscale ou la concurrence déloyale étrangère, commençons par faire respecter par exemple les normes de production instauré au sein de l'Union européenne pour les producteurs par les producteurs mondiaux, Europe, je le disais, meilleure exploitation nos ressources compétitivité voilà donc les 3 principes sur lesquels repose nos plans stratégiques plan que nous avons transmis au gouvernement et que nous appelons à mettre en oeuvre urgemment pour reconstruire notre souveraineté, je vous remercie. Je vous remercie. Donc, la parole est à monsieur Franck ont au nom de la commission des affaires économiques.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, hein, à l'occasion de ce débat, nous voudrions comprendre quelle est la politique de souveraineté du gouvernement en matière d'industrie d'agriculture et de numérique, alors même que les conséquences négatives des délocalisations était perçue par tous depuis des années, les premières études relatives à la dépendance des filières industrielles en même temps, emporter dont été réalisé qu'au moment de la crise liée au Covid 19, quel est donc dans le domaine des industries, la politique de souveraineté du gouvernement les constats ont été faits, il faut désormais en tirer tous les enseignements nécessaires en s'appuyant sur les comités stratégiques de filière, l'État pourrait jouer le rôle d'animateur d'agrégateur par exemple pour faciliter l'achat et le stockage d'un train stratégique sur le fond, nous pensons qu'il faut réinvestir la politique industrielle dans tous ses aspects, dont celui de l'énergie qui est aujourd'hui sans solution à la hauteur des enjeux, nous vous attendons là-dessus monsieur le Ministre des composés, les chaînes de valeur mieux les comprendre, pour les dans l'intérêt national est un impératif, en prenant en compte la totalité du chic de vie des produits que nous consommons des métaux critiques aux produits finaux, nous appelons aussi le gouvernement à développer fortement le recyclage des matières premières levier d'emploi de décarbonation et d'indépendance industrielle pourtant sous-employé l'approvisionnement est aussi un enjeu majeur pour notre agriculture et notre filière agro-agroalimentaire après la désindustrialisation que nous avons connu pendant des décennies, la dégradation forte et constante historique du solde extérieur de notre agriculture témoigner pour de trop nombreux produits de base de moyenne gamme d'une dépendance accrue de la France, la souveraineté alimentaire française et donc aussi en question notre rapport met en évidence, il y a des dépendances forte en matière d'alimentation animale de protéines végétales et d'engrais notamment le cheptel français se réduit d'année en année si l'on veut que l'agriculture française continue à nourrir notre population, il nous faut veiller à la compétitivité de notre production à l'équité des conditions commerciales et un équilibre juste entre protection environnementale et souveraineté alimentaire, quelle est la politique de votre gouvernement pour recouvrer les positions perdues là le 3ème aspect que je veux évoquer est ici la la souveraineté numérique comment appréciez-vous la souveraineté de la France dans le domaine du numérique, Monsieur le Ministre, le Sénat, plaide pour un débat sur l'opportunité de localiser les données à caractère personnel des citoyens et les données sensibles des entreprises sur le territoire de l'Union européenne, dans le cas de de politique de sécurité spécifiques dans l'actualité récente nous rappelle l'urgente nécessité, je pense aux hôpitaux cette localisation des données doit aussi s'accompagner d'une politique de localisation des infrastructures sur le territoire de l'Union Européenne aujourd'hui 80 % des données générées par les internautes français sont hébergés aux États-Unis, il est temps de construire en Europe des infrastructures européennes pour nos usages numériques européens sur terre, hein, nous devons notamment planifie l'implantation de serveur et de centre de données en mer, nous devons doter l'Union européenne d'un réseau brésilien et elle ne dépendant de câbles sous-sous-marins, aujourd'hui détenu par les Gafam et par lesquels transitent entre 96 et 99 % du trafic Internet mondial dans l'espace, nous devons soutenir l'initiative d'une constellation européenne de satellites pour sécuriser nos communications, enfin, nous estimons que les investissements en faveur de la souvent été logiciels doivent être développés, la protection des brevets logiciels français devrait aussi faire l'objet d'une attention particulière est-ce le cas Monsieur le Ministre, si le club européen Gaïa X ne répond pas pour nous à l'impératif de souveraineté des États membres, la stratégie de certification sec nous Claude du gouvernement favorise plutôt les logiciels américains pour assurer notre autonomie technique, il faut développer les investissements en faveur d'une filière européenne du logiciel et de la donner dans les sociétés sont il m'a il immatriculé sur le territoire de l'Union sur tous ces sujets numériques et qui participe toujours plus de la souveraineté nationale tout court, où en est-on, quel est le plan d'action souveraineté numérique de votre gouvernement, je vous remercie. Merci, cher collègue, vous, vous me dites, Monsieur le Ministre, si vous voulez intervenir, allez-y, allez-y. Merci, merci, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente, Prima madame la rapporteure, et monsieur le rapporteur, Montaugé d'abord, merci infiniment à tous les trois, c'est un travail absolument colossale que vous avez engagé que vous avez livré plus de 300 pages et extrêmement utile cartographier les forces et les faiblesses de l'industrie française, ses dépendance par rapport à l'international, en allant extraordinairement dans le détail, vous l'avez dit rapidement dans votre intervention, c'est évidemment extrêmement utile, votre rapport est dense, il est d'extrême qualité et ça ne nuit pas d'extrême quantité également sur l'essentiel de vos préconisations, nous sommes en phase, je le dis d'autant mieux que nombre d'entre elles, le gouvernement a déjà commencé à les mettre en oeuvre, je me suis fait faire un tableau de toutes vos recommandations en mettant du verre quand c'est en cours, du bleu quand merci nous le lançons et en rouge quand on n'est pas d'accord, il y a pas beaucoup de rouge sur ce tableau, on est essentiellement en phase avec vos constats et très largement en phase avec les solutions, j'imagine qu'on aura le temps de l'évoquer ce soir peut-être de petits regrets pour terminer ma première intervention d'abord je vous ai trouvé un peu sévère avec le gouvernement actuel dans quelques titres un peu critique, alors c'est de bonne guerre mais je vous cite par exemple des fragilités de l'industrie dénoncée de longue date mais renforcés à la faveur de naïveté, au pire de de l'inaction des pouvoirs publics, là je dirais que vous avez un ou 2 quinquennats de retard parce que les enjeux de dépendance, on sait, on s'y est attelé depuis 5 ans et la réindustrialisation du pays, je pense qu'elle a commencé il y a 5 ans, on aura sans doute l'occasion d'en reparler : Ce soir, autre petit regret mais là je pense qu'il est plus fondamentale parce qu'au fond le 1er était plus de formes, c'est vous mentionnez assez peu l'attractivité de notre pays qui est désormais la première destination des investissements étrangers depuis 3 ans et je trouve que c'est un atout important qui doit nous permettre d'affirmer que la souveraineté industrielle, c'est à la fois évidemment une force pour avoir une base arrière solide, qui nous permet d'assurer notre suffisance, mais aussi une base arrière qui doit nous permettre de conquérir le monde et j'y crois beaucoup idée sur lequel la protection, c'est pas du protectionnisme, on doit ensemble la la partager, mais sinon vraiment merci et je suis très heureux de pouvoir poursuivre ce débat avec l'ensemble de vos collègues. Merci monsieur le ministre est-ce que l'un des deux rapporteurs ou l'une des deux veut reprendre une minute tout de suite, non seulement on continue le débat donc dans la suite du débat, la parole est maintenant à Daniel Gremillet pour cinq minutes. Ce le président, Monsieur le Ministre, madame, madame la présidente. Madame et monsieur le rapporteur, chers collègues. Effectivement, dans un pays. Il y a 2 enjeux pour qu'vie. Il faut que l'assiette soit pleine pour nourrir l'homme. Mais il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'énergie. Et je voudrais vraiment remercier ce travail qui a été fait. Par tous les trois parce que vous posez vraiment d'une manière très claire la situation dans laquelle se trouve notre économie. Je me au dossier énergétique. Parce qu'il est en train d'impacter d'une manière terrible l'ensemble des secteurs d'activité. Et à cet instant et vous l'avez très bien démontré, il ne faut pas considérer que le dossier énergétique se résume à la crise ukrainienne. Je vais vous donner quelques chiffres, ayant un peu comme d'autres, ce dossier en ligne stratégique de la compétitivité de notre économie, quelles que soient les secteurs d'activité. L'énergie est un élément clé de la compétitivité. Et on vit aussi aujourd'hui, Monsieur le Ministre, encore sur la planification, la stratégie du général De Gaulle sur l'indépendance énergétique sur le nucléaire, les chiffre très clair. Si je remonte à 2009. La France avait un coût énergétique inférieure de 29 % par à l'apport à la moyenne européenne. A 9 % pour les entreprises 30 % si on se prend en considération les ménages. Si on remonte, il y a 10 ans, 2012, on était encore à 27 % de coût inférieur de l'électricité dans notre pays, grâce effectivement la politique qui a été choisi, d'indépendance et je dirais pilotable à travers le nucléaire et l'hydraulique, n'oublions pas qu'on nous avons aussi une énergie hydraulique très compétitive dans notre pays. Et si je reprends. 2018 juste avant la pandémie, là encore, quand je ramène au kW/h produit et acheter lorsqu'on était à 0 euros par kW/h en France, un pays qui est souvent en compétition avec nous sur la relocalisation et la production industrielle. C'est l'Allemagne, et là, effectivement, l'Allemagne était à 0 30, pratiquement le double que nous en 2018.

on était encore avec un Avantage de 38 % en France sur le coup d'électricité par rapport à la moyenne européenne. Mais permettez-moi à cet instant de parler du marché de lundi marché spot. De lundi. Le marché spot de lundi mais notre économie française. Face à 300 euros le mégawatts en France quand il est à 243 euros en Allemagne. Et vous avez compris effectivement que lorsqu'on veut se repositionner en terme de compétitivité lorsqu'on veut remettre en France dans nos territoires, des entreprises de l'activité économique. Tout ce que nous avons construit pendant ces dit pendant ces années nous ont permis effectivement d'avoir des avancées sociales bien plus grande que dans les autres pays de l'Union européenne et si nous rentrons à effectivement dans le détail du coût du travail de l'heure travaillée grâce à cette politique énergétique, notre économie a pu supporter effectivement des avancées sociales qui sont tellement importante pour les femmes et les hommes dans nos territoires. Et si je l'évoque, c'est parce qu'effectivement aujourd'hui cette situation nous amène dans une grande fragilité. C'est une fragilité effectivement qui nous met en situation, et là encore, tous les secteurs d'activité et pas uniquement les roses n'est énergivore qu'on a, on évoque souvent, aujourd'hui, nous avons perdu, activités industrielles très clairement parce que le prix de l'énergie ne permet même plus la production. Mais les entreprises de plus petite taille, nous sommes tous interpellés, vous êtes interpellé sur les territoires effectivement par cette situation, du prix de l'énergie, qui met en situation de précarité et de fragilité pour certaines, d'ailleurs, peut-être même d'arrêt d'activité. Donc le le dossier, il est plus complexe que l'on veut bien le dire, et les mesures qui ont été prises, j'entends Monsieur le Ministre, effectivement, des mesures ont été prises, mais les mesures ont été en terme de conséquences sur l'activité industrielle très limitée puisque, pour la plupart n'ont pas pu bénéficier, et les dernières mesures que vous avez décidé, même si vous avez amélioré le pourcentage par rapport au chiffre affaire exclut encore énormément d'entreprise. Et tout le travail qui a été fait par là, nos collègues de la commission des affaires économiques, qui ambitionne effectivement de repositionner dans nos territoires, une activité économique, on sait tous. Qu'aujourd'hui le prix de l'énergie est un élément déterminant sur le choix d'une entreprise de faire un investissement dans tel pays dans tel territoires.

président, monsieur le président de la République, annonce la création, la nécessité de faire six EPR, c'est pas six c'est 14 qu'il faut tout de suite voir peut-être plus si on a des ambitions industrielles, il y a besoin de se positionner rapidement pour assurer mais il nous faut aussi permettent aujourd'hui d'avoir une activité d'investissements industriel sur la politique énergétique de notre pays pour la la compétitivité, excusez-moi, monsieur le président. Merci, cher collègue, mais si chacun veut pouvoir bénéficier de la réplique, il faut essayer de tenir le temps de parole allez-y monsieur le ministre. Merci monsieur le président merci, Monsieur le Sénateur Gremillet, dont je reconnais là bien volontiers la précision technique, il connaît les chiffres par coeur et il connaît ce marché comme comme personne, et il a bien mis en lumière le fait qu'aujourd'hui on a des contraintes de très court terme lié quand même il faut le dire à la crise en Ukraine mais qui s'ajoute à des enjeux de capacité de moyen terme qui font qu'aujourd'hui effectivement on ne produit pas assez d'électricité en France et nous le regrettons tous et vous le savez, nous y travaillons, est ce qu'on a fait suffisamment aujourd'hui pour protéger l'industrie non, nous y travaillons encore et là dessus je vais être très clair avec vous, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices l'industrie française ne sera pas une victime collatérale de la guerre en Ukraine, nous avons mis en place, vous l'avez dit, un fonds de soutien qui permet quand même un certain nombre d'entreprises, d'en bénéficier, mais vous l'avez dit-il, était insuffisamment flexible et surtout insuffisamment importants dans son ambition, nous en sommes d'entrain de négocier à Bruxelles pour en doubler les plafonds, actuellement de 25 50, nous l'espérons très vite IV. 50 100 millions d'euros et nous souhaitons surtout adapter les critères que vous avez mentionné pour aider les entreprises qui font face à des hausses de facture, vous l'avez vu, nous l'avons vu quand nous sommes allés sur le terrain extrêmement forte. ça ne suffit pas parce que ce fonds, il permet finalement de corriger, a posteriori des pertes qui sont pour la plupart quasiment insurmontable pour les entreprises, l'enjeu majeur, il est aujourd'hui de réduire les coûts, vous l'avez dit, en amont, de réduire les prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz, de ce point de vue là des discussions extrêmement fortes sont engagés à Bruxelles, elles ont pas encore tout à fait atterri mais j'espère vivement qu'elles vont le faire notamment, je l'espère pour plafonner le prix de l'électricité et pour faire ça, aujourd'hui, du fait du déséquilibre de l'électricité nucléaire en France et du fait que, du coup, l'électricité vient en grande partie du gaz allemands on doit baisser le prix du gaz, on est en train d'examiner un dispositif à l'espagnol dont j'aurais peut-être l'occasion de donner les détails un peu plus tard ce soir puisque mon temps cool, mais sachez que nous sommes extrêmement mobilisés au niveau européen, au niveau national et au niveau local pour accompagner nos entreprises, dernier point très important, les entreprises que vous avez sur votre territoire, qui ont des problèmes, envoyez-les nous, on a des CRP les commissaires au redressement et à la productivité, qui sont dans les territoires que vous pouvez mobiliser de manière à ce qu'on puisse aider ces entreprises à renégocier les contrats et on l'espère aussi, hein rebaisser les prix merci. Merci, monsieur le Ministre, une courte réplique monsieur Huré ou même si vous avez dépassé votre temps. Monsieur le Président, je vous promets, je vais vous en donner un peu de temps pour compenser juste Monsieur le Ministre. Que répondez-vous aux entreprises lorsqu'elles vous disent : mais quand le président dit : ne signez pas les contrats, lorsqu'elles sont acculées parce qu'elles sont en rupture de contrat, comment elles vont faire. 2ème question Monsieur le Ministre, elle est, elle est, elle est fort simple : il nous faut accélérer la procédure d'investissement, je regrette que nous n'ayons pas au débat parlementaire, le développement et les choix stratégiques en matière de nucléaire notamment et il y a un point aussi où nous pouvons la et très vite, c'est sur l'hydroélectricité. Merci, la parole est maintenant à notre collègue Franck Menonville pour cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la crise du Covid la guerre en Ukraine le tension d'approvisionnement, la désindustrialisation sont autant de problématiques auxquelles notre pays est confronté, malheureusement, ces phénomènes ne sont que le révélateur d'une fragilité qui s'est installé depuis de nombreuses années dans notre pays le présent rapport dont je veux saluer la qualité, on t'entend tirer les conséquences en proposant 5, plan d'action je voudrais mentionner de chiffres qui illustrent malheureusement notre perte de souveraineté, la gravité de la situation le premier, la part d'industrie dans le PIB a été divisé par 2 depuis 1974. Le second 40 pour 100 de nos intrants industriels sont importés, contre 29 il y a 20 ans notre balance commerciale souffre en effet 900 produits importés génère 80 % du déficit commercial croissant de la France qui devrait franchir cette année plus de 100 milliards d'euros pour 2022, le rapport de nos collègues indique que notre industrie que notre agriculture sont fortement dépendante d'importations critiques telles que les protéines végétales destinées à l'alimentation animale, les métaux ou certaines substances chimiques, la sécurisation de notre accès à ces intrants est crucial, oui à la à l'indépendance, non à la mono-dépendance je voudrais tout d'abord évoqué des traités commerciaux, nous souhaitons une ratification systématique avant l'application des accords commerciaux mixte par les parlements, parce parce que cela renforce le contrôle démocratique et ensuite parce que la ratification permet de prendre en compte l'ensemble des conséquences d'un accord et notamment ses conséquences stratégiques, je crois aussi nécessaire d'aller plus loin en procédant à des évaluations continue dans le temps, par ailleurs, je voudrais revenir, peut être quelques instants sur l'externe, l'ex l'extraterritorialité de certaines législations étrangères qui est préoccupante, le rapport souligne que nous disposons de trop peu d'informations sur les conséquences économiques de ces mesures, des hommes, des amendes faramineuses ont été infligées à des fleurons français et européens menant parfois des acquisitions assez discutable, nous devons protéger nos entreprises car ce n'est pas acceptable qu'une souveraineté étrangère empiète sur celle de la France et de l'Europe, sans capacité de réciprocité notre souveraineté économique passe également par le domaine de l'énergie, la France est condamnée à la dépendance, dans la mesure où elle doit importer des matériaux nécessaires des matériaux nécessaires à la production de son énergie pour autant cette dépendance n'est pas incompatible avec notre souveraineté si nous parvenons à nous approvisionner auprès de sources diversifiées et sur le nucléaire dans l'appart est indispensable dans le mix nucléaire énergétique français est une chance pour notre pays, nous avons malheureusement depuis de nombreuses années, tourne le dos à cette énergies décarbonnées et Douma dont nous avions la pleine maîtrise, il est donc nécessaire aujourd'hui de préserver nos capacités matérielles et de savoir faire les temps qui viennent s'annoncent difficiles, des financements et des investissements conséquents en matière d'énergie nucléaire sont essentielles pour garantir durablement notre souveraineté énergétique, elle devra être renforcée par le développement des énergies renouvelables, autant que possible, mais aussi par la recherche d'économies d'énergie par le la rénovation énergétique par le développement de technologies, plus sobre, mes chers collègues, il nous faut aussi bâtir une souveraineté européenne qui nous permettra de conjuguer transition écologique et défense de nos valeurs et nos intérêts pour développer des solutions efficaces et pérennes, il nous faut travailler de concert avec nos partenaires européens et retrouver la maîtrise de nos dépendances, il nous faut plus vite réformer notre marché européen de l'énergie, il nous faut également revoir notre politique de concurrence pour favoriser l'émergence de leaders mondiaux dans différents domaines tels que l'industrie et l'énergie, nous devons absolument être en mesure de donner les moyens de passer de l'innovation à la réalisation de succès industriel, économique, la France doit absolument réarmer ses capacités industrielles, elle doit maîtriser les technologies de demain, et veiller à ce que ces chaînes de valeur se déploie sur l'ensemble de notre du toi, nous devons tous être conscients que notre modèle social ne peut être financé par cas par un oh que par un haut niveau de performance économique, ce qui fait défaut depuis plusieurs années, l'industrie l'énergie, l'agriculture, même combat, l'innovation et la compétitivité, il est urgent d'agir. Merci, monsieur le Ministre. qui est une des manières d'accompagner au niveau stratégique, les investissements d'avenir, et notamment dans l'innovation, vous l'avez mentionné 54 milliards qui sont destinés, on a élaboré une cartographie très précises, pardon des dépendances dans 5 secteurs stratégiques, l'alimentaire, vous en avez parlé, la santé, l'électronique, les métaux et la chimie l'objectif de France 2030 pour ces 5 secteurs, c'est bien de déployer des fonds qui vont nous permettent de répondre à ces vulnérabilités que vous avez mentionné dans votre intervention, et qui sont très bien documentés dans le rapport, il y a des appels à projets qui sont déjà sortis, près de 300 millions d'euros qui sont disponibles aujourd'hui dans l'alimentation, vous savez que dans l'électronique, c'est plus de 5 milliards qui sont aujourd'hui destinée à renforcer notre notre souveraineté dans l'électronique sur les métaux, vous l'avez mentionné : sujet extrêmement important : le rapport produit par Philippe Varin propose de créer un fonds stratégique qui nous permettra d'investir et de sécuriser des des ressources partout dans le monde voir pourquoi pas, peut être même en France et en Europe et nous y souscrivons et nous y attelons autre point important, vous l'avez mentionné notre capacité à protéger nos fleurons, et c'est vrai que pendant longtemps on a sans doute été un peu trop naïf et vous le savez, puisque nous avons travaillé ensemble sur la loi pacte nous avons renforcé la loi sur les investissements étrangers en France qui fait qu'aujourd'hui les contrôles sont plus systématique ils sont plus larges, il concerne des secteurs plus vaste, un chiffre pour montrer qu'on a accru ses contrôles en 2021 le nombre de contrôles s'est accru de 20 % on a examiné 328 dossiers, dont 124 étaient jugés sensibles 67 d'entre eux ont été délivrées sous conditions et un certain nombre d'entre, on le sait, ont été refusées, on est sur des statistiques finalement assez similaire à ce que font les Américains, merci. Merci. Pas de réplique donc la parole à notre Cowell collègue pardon Joël Labbé. Pour cinq minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Madame et messieurs les rapporteurs. Et chers collègues, la crise du Covid la guerre en Ukraine ont révélé nos vulnérabilités et nos sur les secteurs stratégiques essentiels, les aléas climatiques à venir et l'instabilité internationale nous ne manqueront malheureusement pas devenir aggraver ces problématiques, il est donc essentiel d'agir en urgence pour renforcer notre souveraineté et nous remercions la commission des affaires économiques, notre commission de s'être saisi de ce sujet qui pointe l'insuffisance des réponses politiques actuelles sur ces questions. Nous partageons ainsi une partie des et une partie des éléments présentés par le rapport, dont il est question aujourd'hui comme la faiblesse des ambitions et des actions de l'État sur la relocalisation des filières stratégiques comme aussi la nécessité, développement du recyclage des énergies renouvelables, tout comme l'indépendance face aux Gafam, cependant sur de nombreux axes de ce rapport, nous considérons que la transition vers des systèmes sobre durable et écologique être insuffisamment prise en compte et que les solutions apportées par ce rapport préconisées par ce rapport pérennise certaine dépendance plutôt que de construire une véritable résilience c'est globalement par la sobriété et le développement d'alternatives énergétiques, agricoles d'économie circulaire également que nous pourrons créer des systèmes vertueux est résiliant ah si cela ne vous surprendra pas, nous ne pensons pas que la relance nucléaire soit la solution dans un monde de plus en plus incertain pour assurer notre souveraineté énergétique, je pense à la question de l'approvisionnement en matières premières, la question des risques majeurs en période instable et aussi la question de la gestion des déchets. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir très largement lors des débats, les législatifs à venir nous pensons également que cette réflexion sur la souveraineté, dans un contexte de forte inflation doit toujours aller de Pair avec une réflexion sur la justice sociale, car les tensions que nous connaissons actuellement se répercute aujourd'hui avant tout sur les plus pauvres d'entre nous, voudrais maintenant développer ici plus précisément les questions agricoles, ça ne vous sur prendra pas et la question majeure de la souveraineté alimentaire ici encore nous partageons une partie des recommandations du rapport et encourageant le le gouvernement à s'en saisir, ainsi que la souveraineté de la France doit passer par une forte relocalisation de l'alimentation. En lien notamment avec un soutien renforcé aux projets alimentaires territoriaux, ce sont des outils que nous avons mis en place un soutien accru aux filières de protéines végétales et la mise en place. De la transparence sur l'origine des aliments pour le consommateur, nous soutenons avec force un renforcement du contrôle des produits importés, avec les moyens qui vont avec, si le contrôle ne peut se faire qu'avec des moyens forts. sur le sujet des importations, nous nous devons ici de rappeler le triste anniversaire du CETA entrer en vigueur en septembre 2017 et, à ce jour encore non ratifié par notre assemblée, nous demandons donc au gouvernement, Monsieur le Ministre, d'agir pour mettre un coup d'arrêt à ces accords, aux conséquences délétères nous demandons aussi au gouvernement, à l'inverse de ce que nous propose ce rapport de soutenir la mise en oeuvre ou des objectifs de la stratégie européenne de la ferme à la fourchette, sa remise en cause au nom de la souveraineté serait pour nous une erreur. Stratégique, que ce soit sur la réduction de l'usage des engrais et des pesticides sur l'augmentation des surfaces en agriculture biologique ou sur la biodiversité, il nous faut amorcer d'urgence la transition si on veut véritablement assurer notre souveraineté l'agroécologie est une alternative crédible pour relever les défis climatique et les défis de biodiversité également remettre en cause le pacte Vert au nom de produire toujours plus 7 accentuer la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité, rappelons que les engrais azotés minéraux sont de véritables bombes climatique et que les pesticides qui vont avec son responsable de l'effondrement des pollinisateurs nécessaires à la production agricole, qu'une prise de position forte, monsieur le ministre, une prise de position forte du gouvernement sur son soutien au Pacte Vert européen mais aussi à un règlement pesticides exigeant qui est à l'étude actuellement à l'Europe, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Joël Labbé, alors je pense qu'on va être d'accord pour ne pas être d'accord sur un certain nombre de prises de pas de prise de position que vous avez prise, ça ne vous surprendra pas, donc commençons par les points d'accord quand même le recyclage des matières premières, je pense que c'est essentiel à la fois pour assurer une économie plus durable, plus soutenable, mais aussi renforcer la souveraineté de la France a été dit par un certain nombre d'orateurs mais vous y compris, nous dépendons trop de l'étranger pour des matières premières, extrêmement importante, notamment pour les batteries et vous le savez, dans le règlement, batteries, par exemple, on souhaite qu'à terme 90 % % du lithium inclus dans les batteries fabriquées en Europe ou vendus en Europe, soit du lithium recycler ce qui va à la fois permette de donner un Avantage important l'industrie européenne et il faut le dire de nous protéger contre les importations, parfois un peu sauvage et des dépendances qui le sont trop sur le nucléaire, évidemment, n'est pas du tout d'accord. ça vous surprend pas, je reste et nous restons effectivement éminemment profondément convaincu. Que le nucléaire est une large partie des solutions pour l'indépendance énergétique pour la production d'électricité à bas coûts, ça a été aidé par le sénateur gagner et bas carbone, c'est pas la seule, vous savez que je suis un

moteurs sur les 2 accélérateur qu'on arrivera à terme a littéralement pouvoir rendre la France autonome et surtout accompagner le développement majeur de l'électricité, vous le savez les besoins vont être énorme dans les années qui viennent, vous dites que nous avons insuffisamment protégé les plus démunis, rappelons-nous, quand même, et j'espère, soyons fiers entre nous que l'inflation ne en Europe aujourd'hui les 10 % elle est 2 fois moins à peu près en France, la France est le pays qui a le mieux protéger ces ménages, y compris les ménages les plus démunis contre cette hausse de l'inflation, donc là aussi on sera d'accord pour ne pas être d'accord, et dernier point, je pense que la présidente Sophie Primas s'en souvient, sur le CETA, là on sera vraiment d'accord pour pas être d'accord puisque je l'ai voté, c'est à moi, vous avez raison, il n'a pas été ratifié au Sénat, mais il a été ratifié à l'Assemblée et je faisais partie de la majorité qui l'a voté, Jean-Baptiste Lemoyne, s'en souvient, il était ministre, alors effectivement ça suffit pas, faut qu'il passe ici, mais l'avantage vous l'avez dit, c'est qu'il est en place depuis 5 ans et qu'on peut en en faire un bilan provisoire et que ce bilan, il était extrêmement favorable pour l'économie française si et il n'est pas défavorable pour l'agriculture française. Si Monsieur le Ministre, Joël Labbé une réplique d'une minute. Vous avez encore une minute de répliques, si vous le souhaitez, chers collègues, il y a un micro juste derrière vous. si vous parlez pas dans le micro, c'est compliqué, mais bon, donc on va continuer avec Jean-Baptiste Lemoyne pour six minutes. Bien, monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues, plan reconstruire souveraineté, voilà des mots qui sont à nouveau ancré dans nos politiques publiques singulièrement depuis 2017 et sept heures plan parce que c'est vrai que la main invisible cher Adam Smith, elle résout pas tout, loin de là, c'est quelqu'un qui est très attaché aux libertés économiques qui qui le dit, on dit gouverner c'est prévoir, mais prévoir c'est planifié reconstruire parce que oui, il y a eu des destructions massives, massives, massives dans un certain nombre de secteurs économiques résultant d'ailleurs à la fois de choix faits par les entreprises elles-mêmes dans années 80 90 2000, on se souvient de ce concept, les entreprises sans usine voilà à quoi ça conduit et puis aussi parfois l'état qui s'est retiré, hélas à mauvais escient et puis souveraineté parce que oui, il est temps de reprendre le contrôle de notre destin et ça passe, ça a été dit par la rapporteure et par monsieur villes par une souveraineté recouvrée, tant au niveau national qu'au niveau européen, il ne faut pas les opposer, je me réjouis que les travaux conduits par notre assemblée et la commission des affaires économiques et puis aboutir à cette boussole avec du véritable feuille de route thématiques et ses objectifs, nous les partageons au groupe RDPI, c'est le fil rouge d'ailleurs que tire le président de la République depuis 2017 jouit d'une souveraineté d'une indépendance accrue et l'idée c'est que on reprenne ce contrôle, donc en tant que Français et bien sûr, mais, mais aussi en européen et pas en solitaire, comme ça a été fait de de l'autre côté de la Manche et et l'idée c'est qu'on soit pas des objets de l'histoire qui s'écrit, mais bien des sujets qui maîtrisons notre avenir alors rebâtir la souveraineté économique, l'indépendance industrielle, ça a été au coeur des politiques conduites depuis 2017, les résultats sont là, tangibles, réelles, je pense aux baisses d'impôts à Liesse et qui va se poursuivre avec la baisse de la CVAE ça fait que la France, elle est le premier états de lieux en termes d'investissements Directs étrangers désormais on ouvre plus d'usines qu'on enferme dans ce pays et de l'emploi industriel et recréer, et puis il y a également l'État qui se réarme 7 heures avec France relance avec France 2000 on le voit un exemple très concret face à la concurrence sino-américaines dans tout ce qui est micro-électronique, hé bien le site, estime au micro électronique à Crolles, en Isère accueillera une nouvelle usine de semi-conducteurs, c'est 1000 emplois supplémentaires d'ici 4 ans un énorme investissement industriel de ces dernières années je reprends entre guillemets ou un affichage politique pour reprendre des termes inutilement taquin du rapport, ce sont de véritables mesures qui conduiront à une réindustrialisation massive de la France avec l'objectif d'ailleurs à 2030, hé bien de retrouver le niveau d'industrialisation manufacturière de 12 % on est tombé plutôt autour de neuf avec 450000 emplois à la clé et puis au niveau européen, le réveil a sonné également, il serait d'ailleurs absurde que l'Europe qui a, qui est né à travers le le le la construction économique se fasse dicter sa loi qu'elle renonce une puissance économique qui s'assume comme telle, alors comment hé bien en forgeant nos propres standards, bref en évitant d'être les idiots utiles du village global et pour cela, un certain nombre de révolution copernicienne ont été menés, doivent se poursuivre, avec à nouveau des politiques industrielles au niveau européen, souvenez-vous, c'était voilà, il y a quelques années encore inimaginable d'avoir ces ces, ces coopérations poussé à ce niveau-là, en nous dotant aussi de nouvelles règles en matière de politique commerciale pour ne pas être ouvert aux 4 vents sans réciprocité réciprocité c'est un terme d'ailleurs qui était devenu un gros mot effectivement du côté de Bruxelles, hé bien, c'est un terme qu'on a remis au goût du jour avec les clauses miroirs qui permettent de garantir la réciprocité des normes environnementales avec nos partenaires commerciaux avec l'instrument de réciprocité sur les marchés publics, les fameuses adopté après plus de 10 ans de négociations qui remet de la concurrence équitable entre les entreprises européennes et les entreprises étrangères alors pour l'avenir les les sénateurs du groupe RDPI, seront heureux d'être au rendez-vous sur bon nombre de recommandations issues du rapport en matière de souveraineté de l'approvisionnement oui consolider notre effort en matière

voilà peut-être de travailler des ajustements, le ministre a rappelé récemment, cette stratégie, elle a été adopté, 6 mois avant la guerre, en Ukraine et un débat peut se nouer au niveau européen, là dessus, et puis oui, en matière de souveraineté des infrastructures énergétiques numérique avec sa souveraineté nucléaire que nous devons maintenir consolider souveraineté des métiers et des compétences, quand le 4ème chantier oui, avec un financement pérenne ambitieux de l'apprentissage, je rappelle les résultats obtenus et et le 1000000 de contrat sera atteint grâce notamment à 5 milliards d'euros qui sont prévues dans dans le prochain budget et puis en matière de souveraineté commerciale, ça a été dit, oui, 3 fois oui au au déploiement de de ces clauses miroirs et je terminerais avec la souveraineté des entreprises qui est le 5ème chantier 5ème feuille de route, évoquée par les rapporteurs, je crois que il est important d'avoir une véritable démarche d'Intelligence économique et avec Marie-Noëlle Lienemann, c'est un sujet qui nous est cher, sur lequel nous pensons que nous pouvons, nous, Français, muscler notre jeu écrit peut être un véritable programme national d'Intelligence économique qui implique les pouvoirs publics, les entreprises, bref pour mieux assurer la défense et la promotion de nos intérêts économiques, industriels et scientifiques c'est fait assez systématiquement outre-Atlantique je crois qu'on gagnerait, là aussi, hé bien à regarder ça de plus près, voilà un autre travail transpartisan qui pourrait être utile et aboutir la prise de conscience, on l'a vu, elle est là, les actions, elles ont débuté, il nous faut maintenant je dirais maintenir l'effort et et accélérer même compte tenu du contexte, il y avait les les 12 travaux d'Hercule, il y a désormais les 5 plans de souveraineté du Sénat, hé bien je le dis à la Commission comme au ministre, nous serons à vos côtés pour avancer, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Monsieur le président, merci Monsieur le Ministre pour pour cette intervention je me je concentrerai peut-être ma réponse sur votre dernier point puisque c'est celui sur lequel vous avez jugé, je pense que c'est utile qu'on pourrait s'améliorer sur les enjeux d'Intelligence économique et dans une capacité à préserver la souveraineté de nos entreprises, alors il y a des choses qui existent, vous le savez, vous avez étudié ce sujet de prêt avec votre collègue, j'aimerais quand même les rappeler, donc il y a des actions préventives, vous savez qu'il y a un service à Bercy, qui s'appelle le service de l'information stratégique et de sécurité économique, le six qui fait un suivi des vulnérabilités des mouvements de capitaux, des investissements étrangers, de manière à assurer une veille stratégique éventuellement d'alerter, vous le savez aussi, c'est assez récent que en cas de montée au capital ou même d'intérêt marqué d'investisseurs étrangers vis à vis d'entreprise que nous jugeons stratégique nous pouvons intervenir, nous avons créé un fonds qui s'appelle le Front French Tech souveraineté 2030, qui nous permet d'intervenir et de monter au capital, enfin je l'ai dit tout à l'heure, la procédure investissements étrangers en France, a été élargie et renforcée pour autant, on peut sans doute faire mieux, vous l'avez dit, je suis prêt à le reconnaître, monsieur le Ministre, je sais que ce sujet vous tient à coeur avec votre collègue et donc moi je suis prêt à suivre effectivement tous les efforts que vous mènerez ici pour mieux structurer notre approche n'oublions pas évidemment que la limite est fine entre la naïveté qui a parfois peut-être un peu trop régner chez nous et le protectionnisme, auquel je suis moi-même, extrêmement opposés mais cette ligne fine entre les deux elle existe et je suis sûr que nous pouvons la dessiner ensemble merci. merci beaucoup monsieur le président, merci Monsieur le Ministre, pour cette réaction, je pense que sur l'Intelligence économique, j'ai bien en tête tout ce qui se fait à Bercy je pense qu'il faut une véritable dynamique interministérielle fait ça concerne c'est très transversal, effectivement, on le voit bien, Défense, Affaires étrangères et etc, et, et et voilà et donc donner une impulsion supplémentaire en terme en terme voilà de conduite de cette politique, mais merci en tout cas pour votre ouverture à ce que le travail se poursuivent, de cette façon-là, merci. Merci, cher collègue, la parole est désormais à notre collègue Florence Blain Trix content. Pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes ici pour interpeller le gouvernement sur la base du travail au sein de notre commission des affaires économiques, pour reconstruire la souveraineté économique en France et en Europe, ça me donne l'occasion tout d'abord de souligner la qualité vraiment de la contribution de nos rapporteurs la pandémie a conduit un retour au 1er plan de la souveraineté économique, il ne s'agit pas d'une souveraineté qui s'opposeraient aux échanges et à l'ouverture, il s'agit de réduire nos dépendance vis-à-vis des productions essentiel, l'enjeu est de définir les biens et les services stratégiques et de mettre en oeuvre une méthode une méthode pour recouvrer l'indépendance nécessaire parmi les secteurs essentiels : le numérique est particulièrement important, alors que notre économie, notre société ont été profondément transformés par le numérique, la question de la souveraineté Méric s'est posé posé avec acuité et je travaille d'ailleurs sur le sujet avec notre collègue Catherine Morin-Desailly qui a été peut le dire, une pionnière une pionnière en France en la matière, nous avons proposé à la Commission européenne différentes résolutions visant la la régulation des marchés, des grandes plateformes mais aussi l'amélioration du projet de boussole numérique qui traduit les ambitions numériques et de l'Union européenne pour 2030 à ces enjeux économiques s'ajoutent les enjeux de sécurité mais également des enjeux éthiques et sociétaux la dépendance aux acteurs américains et chinois n'est pas seulement catastrophique d'un point de vue économique elle est incompatible avec nos valeurs et la vision de la démocratie que nous portons pour assurer notre souveraineté, il faut d'abord sécuriser les approvisionnements le rapport articule justement action des autorités européennes et françaises, la démonstration est sans équivoque : nous avons besoin de plus d'Europe mieux ciblée, active et efficace et cela a déjà été évoquée dans la négociation des accords commerciaux internationaux, les institutions européennes doivent mieux protéger et promouvoir les productions et les réalisations européennes par sa capacité de financement Direct via les fonds spécialisés ou indirecte, via les capacités de près les institutions européennes, en coordination avec les États membres doivent contribuer à l'émergence d'écosystèmes industriel et sectoriel européen d'avenir, comme cela est mis en place pour la défense, nous avons besoin d'un vrai système de Claude européen souverain d'un Gaïa X qui ne soit pas sous influence et d'un euro numérique qui ne soit pas géré par Amazon, aujourd'hui, la confusion règne voulons-nous vraiment nous donner les moyens de faire sans les Gafam et comment votre gouvernement contre-t-il agir pour limiter notre dépendance aux acteurs extra-européen pour recouvrer autonomie stratégique et souveraineté, l'investissement dans les compétences est essentiel n'est de richesse que d'hommes, écrivait Bodin et nous devons tenir compte des difficultés de recrutement du secteur et adapter nos formations en matière de numérique cela à tous les niveaux, que ce soit au niveau du bac pro ou du BTS du bahuter des diplômes d'ingénieur et, bien entendu, en ayant recours à l'apprentissage, c'est très important et, à cet égard je suis particulièrement inquiète quand même de la baisse étayée par les classements internationaux du niveau en mathématiques de nos élèves qui sera particulièrement préjudiciable pour le le secteur du numérique, il s'agit, en matière de formation de repenser l'offre de formation dans les domaines du numérique dans les secteurs stratégiques de de ma le Cloud l'Intelligence artificielle, l'informatique quantique et comment le gouvernement compte-t-il agir afin de permettre au secteur du mérite d'être doté du capital humain essentiel à son développement. Par ailleurs, la puissance publique doit elle aussi montrer l'exemple, je pense ici à la plateforme des données de santé au logiciel utilisé dans l'éducation nationale ou dans les administrations publiques, enfin le rapport insiste sur le caractère hautement stratégique et les interactions entre les infrastructures énergétiques et numérique, je veux insister sur la complémentarité essentielle entre ces 2 domaines d'activités : les activités numériques et et Digital nos entreprises en général et en particulier nos collectivités ont besoin d'un approvisionnement électrique stable sur avec une visibilité en termes de prix donc avec le conflit en Europe orientale, l'indépendance énergétique redevient un sujet d'actualité sans hein d'indépendance énergétique, il ne peut y avoir de politique économique, industrielle, souveraine et surtout de réindustrialisation, donc en France et en Europe nous devons programmer les investissements pour organiser la transition énergétique vers les énergies décarbonnées nécessaire et au-delà de l'urgence, il faut répondre aux besoins de moyen et de long terme et à cet égard la question du projet national pour EDF, désormais 100 % public sera centrale et devra être publiquement des pâtes débattu au Parlement et dans le pays et donc le rapport qui nous est soumis, trace un chemin, il nous faut désormais une volonté, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice la triste compta merci pour pour vos remarques, vous avez vous aussi couvert beaucoup de terrain, je vais peut-être me concentrer sur le numérique, qui est un sujet qui vous est cher et auquel j'ai relativement peu répondu : vous avez raison, moi je préférerais qu'on ait un souverain français ou européen, on n'a pas à ce stade encore, j'espère que ça viendra de fournisseur non américain, il faut le dire, Google, Microsoft et quelques autres sont son seul sur le marché, on y travaille, j'espère qu'on pourra faire émerger un champion mais en attendant, vous le savez aussi dans le cadre du projet Cloud souverain auquel Bruno Lemaire notamment, mais mon collègue Jean-Noël Barrot également sont très attachés, on a une procédure de Nancy qui va permettre de faire une véritable muraille de Chine entre ce qui sera fait en Europe, protection des données, conservation des données nationalités des employés pour éviter l'extraterritorialité américaine et cetera, et cetera qui permettra de développer ce que la de souverain dans un 1er temps sans doute avec des fournisseurs non européens mais de logique dans une logique extrêmement isolés, isolés, donc j'espère que vous en serez rassurée en tout cas, nous en sommes extrêmement conscients, vous avez beaucoup parlé d'apprentissage et notamment de l'apprentissage des mathématiques, je pense qu'on est tous convaincus qu'on a besoin de plus d'ingénieurs et d'ingénieurs en France, moi ce sera un de mes combats, j'y reviendrai peut-être dans mes remarques conclusives, la formation, l'apprentissage, notre capacité à former des ingénieurs et je le répète et des ingénieurs sera un naissance un facteur essentiel du succès de l'industrie française, merci madame la sénatrice. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, allez-y. Merci, monsieur le Ministre de votre réponse, je ne suis pas complètement convaincu sur votre vos modalités de Claude souverain et je pense vraiment qu'il faut promouvoir et faire confiance aux acteurs français et européens en les matières en la matière, on a vraiment perdu des pépites qui sont partis à l'étranger et voilà, je pense qu'il y a vraiment une action renforcée en la matière, je vous remercie. Merci, la parole est désormais à notre collègue Fabien Gay. C'est le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au début des années 90, les libéraux ont pensé que c'était la fin de l'histoire, le capitalisme était triomphant tout devait être gérée par le marché libre et non faussée la libéralisation des secteurs de l'énergie, des transports, des communications, à les faire baisser les prix et permettent d'innover et l'État, surtout ne devait être ni interventionniste ni protectionniste, ni même régulateur plus aucune limite dans les profits dans l'exploitation du vivant et de la nature ni frontières et ni barrières douanières, la grande compétition internationale, allez faire des gagnants et quelques perdants mais le tout était de se spécialiser dans les produits finis et à haute valeur ajoutée, fidèle au précepte de Ricardo, pire, on pensait que l'idéal, c'était une France sans usines comme Serge Tchuruk, alors PDG d'Alcatel qui, déclaré qu'il souhaitait une entreprise sans usine pendant 30 ans, nous avons assisté à une dizaine de Russes réalisation du pays, pensant qu'une France des services nous placerait au 1er rang des grands gagnants, mais la crise sanitaire et la crise énergétique nous ont ramener à une triste réalité nous avons manqué de tout, et lorsque l'usine du monde, la Chine a été à l'arrêt, nous sommes mis en difficulté surtout même les biens de première consommation de première nécessité, notre affaiblissement n'est pas qu'industriel, il agricoles, énergétiques, mais il est surtout dans toute la chaîne de valeur dans l'industrie, lorsqu'on ne maîtrise plus toute la chaîne de valeur que l'on ne dépendent de pièces fabriquées à l'de l'autre côté de la planète pour faire par exemple moteur nous nous mettons en difficulté pour construire nos propres voitures cette désindustrialisation ce déclin de nos savoir-faire de nos compétences, c'est un drame que nous sommes auto-infligée la croyance dans la dérégulation de l'économie nous a conduit à l'affaiblissement à renforcer notre dépendance envers l'extérieur et quand on fait cela, on concède chaque fois un peu plus de souveraineté, prenons le cas d'une économie dans laquelle nous avions tout pour avoir un potentiel français le numérique après la privatisation de France Télécom, la France a vendu Alcatel-Lucent un Nokia, achevant ainsi de démanteler le Patrimoine industriel nécessaire à cette innovation technologique aujourd'hui, nous continuons à reproduire les mêmes erreurs, parlons du tant attendu Health Data hub, cette plateforme centralisée des données de santé française aurait pu être une aubaine pour nos développeurs français du digital à-t-on de choisi l'un d'entre eux pour développer le projet comme OVH, par exemple, non c'est à Microsoft qu'il a été attribué, sans même passer par un appel d'offres, voyez le message que nous envoyons à nos entreprises françaises sur des opportunités exceptionnelles, voyons les dégâts que nous infligeons à notre propre souveraineté, il nous faut que par exemple, comme le propose ma collègue Marine Waldman, un véritable programme national d'Intelligence économique sur l'approvisionnement en même temps en matière de souveraineté alimentaire faisant le bilan de tout, c'est très très de libre échange CETA JEFTA Merco sourd, Singapour et encore récemment, la Nouvelle-Zélande, c'est le choix d'un modèle dans lequel on importe des produits dopé à des substances interdites au sein de notre Union européenne, c'est le choix de dire à nos filières agricoles françaises, européennes, que tous les efforts qu'on leur demande ne paieront pas devant les consommateurs puisqu'ils achèteront du moins cher, du moins bon et du venus ailleurs, outre le non-sens économique et écologique de ces traités quand nous parlons de souveraineté économique gardons en tête que la politique commerciale de la Commission européenne n'écarte toujours pas la possibilité que des investisseurs puissent signé un État devant un tribunal de justice cet aspect du CETA, dont nous, et nous espérons un jour débattre en est le parfait exemple criant le tout libéral le marché dérégulé n'a rempli aucune de ses promesses, pire, il nous a fait décliner la crise de l'énergie, nous en apporte un nouvel exemple l'affaiblissement d'EDF au profit d'opérateurs privés qui se sont enrichis sans investir dans la production, les tergiversations du gouvernement sur le nucléaire, nous ont conduit précisément à l'état du parc nucléaire que nous connaissons aujourd'hui, et à la perte de notre souveraineté nous énergétique mais il n'y a pas de fatalité, nous pouvons reprend le contrôle de notre économie en relocalisant, en conditionnant toutes les aides publiques à la sauvegarde de l'emploi et de l'industrie et en fait en sortant des secteurs stratégiques du secteur marchand, comme le NPA d'énergie et enfin sur des grands domaines énergie numérique spatiale Télécom santé et produits pharmaceutiques bâtissons non pas dans la compétition, mais dans la coopération et la solidarité des grands champions européens permettant de réussir la transition énergétique et de remplir notre devoir de souveraineté économique européenne, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur gay bon une partie des des reproches que vous adressez, je les prends et je pense qu'on peut les prendre en collectivement, ça fait une trentaine d'années, qui ont désindustrialisé la France, j'allais dire qu'désindustrialisé la France parce que cette tendance à la baisse s'est inversée, on doit maintenant accélérer depuis 5 ans, elle s'est inversée, on a créé des usines, 3 fois plus d'usines en France en 2021, qu'on n'en détruisaient on a créé 50000 emplois dans l'industrie, c'est insuffisant, mais ce sont quand même des créations d'emplois depuis 5 ans, il va falloir continuer accélérer évidemment, je ne serais pas d'accord avec vous, surtout moi je souhaite pas forcément jeter le bébé de la concurrence avec l'eau du bain du libéralisme exacerbé, je ne suis pas un libéral sauvage je pense que la concurrence a des vertus, vous avez parlé d'Orange, c'est aujourd'hui une entreprise nationale qui est un grand champion qui est reconnu dans le monde entier et qui fait quand même que grâce à la concurrence, on paye aujourd'hui nos téléphones en Europe nos abonnements, y compris à des données qui sont extrêmement utiles, 5 fois moins cher qu'on le fait aux États-Unis, le soit disant pays du libre-échange et du libre-marché, donc la concurrence, elle a des vertus maintenant là où vous avez raison, c'est que le mythe du faiblesse, la fameuse usine sans usine de l'ancien patron de d'Alcatel, que vous avez bien voulu citer, c'était une chimère et nous avons besoin effectivement à la fois pour des raisons économiques, mais j'en suis convaincu aussi pour des raisons politiques, d'une conne d'une colonne vertébrale industrielle dans nos territoires, moi ma feuille de route, aller simple, on m'a demandé de réindustrialiser dans les territoires partout et pour tous et pour toutes, un enjeu de formation extrêmement important, un enjeu d'attractivité du territoire, un enjeu de travail en collaboration avec l'ensemble des élus locaux, régionaux et nationaux et 54 milliards quand même, c'est pas rien de France 2030, qui vont nous permettre de le faire, donc je pense qu'on est aligné sur les objectifs, on sera peut être pas forcément alignée sur toutes les solutions, mais sachez qu'en tout cas je pense que sur l'industrie, on a à peu près tous le même maillot que j'espère qu'on jouera dans le même sens, merci. C'est monsieur le président, Monsieur le Ministre, je ne sais pas si on a le même maillot ni la même passion pour le libéralisme, ça c'est sûr, mais oui, il faut faire quand même un peu le bilan de toutes ces libéralisations et de toutes ces ventes forcées, vous le dites, on industrialise très bien, mais le président Macron il a été au coeur de la vente de Technip de Nokia, de General Electric dans un certain nombre de domaines stratégiques qui nous manque encore aujourd'hui, pardonnez-moi et je ne lis pas les efforts qui sont faits depuis le plan de relance, France 2030, mais on a, on peine quand même avoir les effets réels aujourd'hui dans les territoires, vous nous dites, on veut créer de l'emploi industriel pour l'instant, on continue à en perdre et des grandes entreprises et nous les mettons en difficulté sur la question énergétique par exemple Duralex par exemple l'Arc International qui vont plus pouvoir produire parce qu'aujourd'hui la facture électrique du fait de la libéralisation de ce secteur va peser trop lourd et ils vont préférer mettre en réalité aujourd'hui un certain nombre de salariés au chômage partiel, voilà la triste réalité du bilan, la libéralisation d'un certain nombre de domaines économiques, je vous remercie. Merci, la parole maintenant à notre collègue Catherine Morin-Desailly pour quatre minutes.

et je m'en réjouis, ont été, je le dis avec humilité, une des premières à avoir été sur la perte de souveraineté qui menaçait l'Europe dès 2013, dans un rapport, l'Union européenne que Lily du monde numérique aujourd'hui on en parle et c'est fort fort heureux, le numérique n'est pas une industrie, mais toutes les industries, toute l'activité humaine étant amené à se numériser notre groupe ne cesse de dire qu'il y a là un enjeu stratégique pour le devenir de nos sociétés Internet est désormais un terrain d'affrontement Mondia dont l'enjeu et la domination du monde par l'économie et la connaissance or jusque-là, les gouvernants ont laissé des acteurs extra-européens s'imposer sur le marché et constituer des menaces à terme systémique pour notre économie et des risques pour les États dans leurs fonctions régaliennes risque d'ingérence, de manipulation de la part de pays étrangers cyber attaques en tout genre désinformation gangrénant les réseaux. Sociaux, il aura fallu l'accélération de la numérisation notre économie avec la crise sanitaire et le confinement pour prendre conscience du besoin de développer nos infrastructures, en particulier celles liées au Claude Le Claude c'est des câbles, des Data centers des serveurs, mais aussi des briques logicielles tout cela représente un énorme marché des milliers d'emplois et tout se segments à très forte valeur ajoutée est aujourd'hui cannibalisé par des entreprises étrangères que nous encourageons même nous privant de faire émerger un écosystème européen indépendant alors du sursis au sursaut oui en effet il est plus qu'urgent de reprendre en main notre destin numérique du nom d'un autre de mes rapports portant sur l'urgence de la formation et de pousser tous les curseurs l'Union a adopté le Digital Markets Act et le Digital savez ces actes texte règlement sur les marchés, services numériques permettant enfin une régulation dont le développement d'un marché aux coalitions plus équitable et loyale, c'est très bien mais il faut aussi et surtout mener une politique industrielle du multi-Cloud pour rééquilibrer les rapports de force et protéger la donner, devenu un actif stratégique majeur sécuriser le Patrimoine économique et industriel dans le Cloud, c'est absolument cela apparaît peu hélas dans le plan d'action, horizon 2030 appeler boussole numérique dont on ne sait comment il sera financé et quelles seront les modalités permettant d'atteindre les objectifs de reconquête d'autonomie il y a aussi les plans de relance, comme les Américains, les Russes ou les Chinois ont su le faire pour eux-mêmes, il faut faire de la commande publique le 1er levier pour boosté la compétitivité du Cloud français et européen et cesser d'acheter des technologies étrangères, quand leur marché en plus nous sont fermés depuis 2013, je plaide pour un Small Business act à la française et un bail acte pour soutenir et développer un tissu d'entreprises à l'origine de technologies innovantes aux solutions de Claude sécurisée et responsable côté environnemental, cela suppose une doctrine de responsabilité Monsieur le Ministre, inexistante aujourd'hui au sein de la 10 num et un rôle proactif de la part de l'État actionnaire, pour cela il faut structurer le dialogue entre ses services et l'écosystème français des PMI et ETI du Claude, elles sont en train de se faire, nous avons noté le récent changement de discours de la part de Bruno Lemaire on aurait ont enfin fini avec le dénigrement de nos propres entreprises cultivée par l'ancien secrétaire d'État au Numérique Cédric O, dont la stratégie à contretemps du Cloud dit de confiance a consisté à confier la gestion des données les plus sensibles, la nation au géant américain, et ce en l'absence d'accord européen de transfert de de donner vers les États-Unis, c'est le cas de la plateforme des données santé évoqué ici la confier à Microsoft, alors que derrière, les questions de recherche, c'est toute l'économie de la santé, le secteur assurantiel et pris prudentielles qui est en jeu, demain le récit selon lequel nous aurions 3 décennies de retard et insupportable et inexact dans quel autre secteur industriel entretien ton ainsi l'image que les Français sont mauvais aujourd'hui nos entreprises se rebiffe et se mobilisent, elles ont bien raison, récemment, Hexatrust a remis à Jean-Noël Barrot un manifeste que j'ai soutenu plaît tant pour ces mesures cria au groupement des entreprises européennes du Cloud récemment réunis à Bruxelles, porte les mêmes revendications, alors oui, madame la rapporteure du sursis au sursaut Monsieur le Ministre, ne croyez-vous pas qu'il est vraiment temps de passer du slogan de la Start-Up nation au plan d'action de l'infrastructure nationale je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Merci madame la sénatrice Morin-Desailly. La Start-Up nation est-ce que c'est si grave, est ce que c'est si mal aujourd'hui, c'est quand même un 1000000 d'employer en France. Donc c'est peut-être pas la réponse à tout, mais j'ai, j'espère quand même ensemble, on peut reconnaître que depuis une dizaine d'années, d'ailleurs ça datait un peu d'avant nous, puisque ça a été lancée dans le mandat précédent la French Tech est un vrai succès, ça ne résout pas tous les problèmes, vous l'avez mentionné clin devra je pense que j'ai répondu tout à l'heure sur ce sujet particulier en attendant qu'on ait un champion français, certains ont essayé, ils n'ont pas réussi, on a mis en place les murailles de Chine qui nous permettent de protéger les données et d'éviter qu'elle puisse être captée par un Américain, avec un certain nombre de remarques, je vois que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pourrez sans doute y répondre de Annecy qui permettent d'assurer la protection mais la French Tech, aujourd'hui c'est quand même 8 milliards d'euros de de de fonds levés, cette année, 10 fois plus qu'en 2017, je le répète, c'est un 1000000 d'emplois c'est des Start-Up industriel dans lequel nous souhaitons investir avec un objectif extrêmement ambitieux 1500 Start-Up industrielles avec 100 nouvelle usines parents que nous souhaitons construire, j'en ai rencontré un certain nombre, elles sont extrêmement dynamique, elles vont irriguer nos territoires soyons fier de la French Tech, soyons fiers de la Start-Up nation ça ne résoudra pas tout, mais aujourd'hui c'est un moteur très clair sur les PME, vous avez raison, il y a pas de Small Business ni à la française, ni à l'européenne, les achats, pour moi, c'est un élément ex-sensuelle de ma mission, j'y reviendrai dans mes remarques terminal je voudrais quand même rappeler que dans le cadre de France 2030 54 milliards 50 % de ces fonds doivent aller à des PME et aujourd'hui à tous les à AP qu'on lance, on a des PME qui réponde, qui réponde avec beaucoup d'énergie à ses appels à projets et donc on est très heureux de pouvoir aider nos PME françaises, elle aussi, à innover, à épouser les révolutions technologiques qu'on soit pousser dans le cas de France 2030. Merci monsieur le ministre, chers collègues, allez-y. Bien entendu l'instar, toutes les jeunes, ce sont des emplois mais à quoi bon, si c'est pour que ces Start-Up qu'on a aidé au démarrage soit racheté assez rapidement, faute de plan de développement et d'infrastructures pour pouvoir les les conserver, donc si on a assez peu d'agents d'investir, investir autant que ça soit éminemment stratégique, je l'ai dit, les enjeux sont devenus politique et géopolitique aujourd'hui monsieur le Ministre, et vous aurez beau construire toutes les murailles de Chine que vous voudrez, la législation américaine date quatre font que de toute façon, en l'absence de preuves Sicile invalidé il y a plusieurs mois, nous sommes sur la jurisprudence Shrek deux hé bien nos données les plus stratégiques les plus sensibles sont fragilisés, quoi qu'on en dise, quoi que fasse l'Annecy, je vous le dis tous les meilleurs spécialistes, les meilleurs juristes qui détecte la façon d'où ça s'est passé le dix aujourd'hui, donc c'est un pis-aller que d'acheter des licences coûteuses pour acheter des nouvelles des technologies européennes investissons plutôt dans nos entreprises qui existent, on peut acheter des briques de logiciels et construire progressivement progressivement cet écosystème dont nous avait nous avons tant besoin aujourd'hui, voilà pourquoi c'est dans l'infrastructure de Nelson aujourd'hui qu'il faut vraiment investir je, je vous le dis, et vous avez en France justement toutes ces PME en Europe ces ETI qui se sont très éloigné des préoccupations de la DGE et qui demande à vous rencontrer, qui demande à jouer leur partition dans cet enjeu éminemment stratégique, aujourd'hui, je crois qu'on a plus le droit de se tromper aujourd'hui et la loi FISA et là elle nous rappelle que le plein de confiance, c'est un faux nez pour la souveraineté.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, amis mais Naples et messieurs, pardon, les rapporteurs, mes chers collègues, tout d'abord je voudrais féliciter les rapporteurs pour ses propositions précises, la qualité du travail de notre assemblée, est à la hauteur des défis que nous traversons, pourvu que les actes suivent les rapports Monsieur le Ministre, mais veut nos enfants, je voudrais rappeler que le terme souveraineté nous vient du latin super U, ce qui signifie dessus pour votre gouvernement, Monsieur le Ministre, c'est l'Union européenne qui est super russe le dessus de tout et c'est là, si j'ose dire que le bas blesse, car pour notre Constitution la souveraineté est nationale, elle appartient au peuple français la souveraineté signifie liberté autonomie et protection, c'est pourquoi elle ne se partage pas, elle ne souffre d'aucune concurrence le présent rapport aurait donc pu s'appeler reconstruire la souveraineté économique française, sa souveraineté nationale, n'empêche pas une coopération européenne dans de nombreux domaines et je l'appelle même de mes voeux, mais elles restent incompatibles avec le projet fédéraliste européen depuis des décennies, les gagnants de la mondialisation ridiculiser jusqu'à l'usage de ce terme de souveraineté sans prendre la mesure de l'effondrement français qui étaient en cours, désindustrialisation délocalisation détresse paysanne, concurrence déloyale, dumping social recours massif aux travailleurs détachés, résultat : nous avons perdu tant de nos savoir-faire et de nos outils de production que nous sommes dépendants de l'étranger, le déficit commercial de la France a atteint 71 milliards d'euros au 1er semestre 2022, un record absolu extrêmement inquiétant, les crises révèlent au grand jour, mot dépendance c'est la cigale et la fourmi, à l'échelle d'une nation, nous avons été incapables de prévoir l'orage durant le beau temps, les crises nous font découvrir que les États ne sont pas automatiquement ni éternellement des partenaires bien intentionnés le présent rapport évoque l'importance des réformes structurelles, sans questionner notre soumission juridique à l'Union européenne depuis 30 ans, sous couvert de libéralisme, les gouvernements français ont cessé de défendre et de planifier les intérêts régaliens à l'État, stratège, a succédé l'État obèse voulant s'occuper de tout, est désormais trop impôts impotente pour investir dans les secteurs clés, lundi, le 1er ministre a annoncé vouloir reconquérir notre souveraineté c'est l'aveu que notre souveraineté était perdue et que l'intérêt national n'était plus au coeur de votre politique, c'est 5 plans sur la souveraineté économique proposé par mes collègues ne peuvent être décoré les du rapport sénatorial de cette semaine sur la souveraineté alimentaire, notre pays est passé de 2ème à 5ème exportateur mondial en 20 ans et nous importons désormais 50 % des denrées alimentaires consommés dans notre pays aujourd'hui, les mécanismes de l'Union européenne en n'empêche pas les hyperpuissance étatiques, comme la Chine et les pays du Golfe de racheter des pans entiers de notre territoire, la commission n'est pas non plus crédible pour nous défendre face à la voracité des Gafam, il faut le retour de ne pouvoir régalien pleinement souverain pour endiguer les vues des hyperpuissance privée sur nos domaines personnel sur nos données pardon personnel et nos vies, le pilotage de l'industrie ne devrait pas se faire depuis un ministère délégué mais d'un super ministère dédié puisse la crise Monsieur le Ministre, nous permettre de retrouver un état stratège audacieux et courageux, une vision véritable indispensable à la reconquête de la souveraineté économique de notre pays. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Si Monsieur le président, Monsieur le Sénateur Ravier, ça c'est sûr que si il y a bien un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, c'est le rapport à l'Union européenne, je reste, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagé politique convaincus engagé en politique, il a maintenant un peu plus de 5 ans que l'Europe fait partie des solutions et pas des problèmes, elle est pas parfaite, elle a beaucoup évolué depuis 5 ans, mais si vous aviez été au pouvoir depuis 30 ans, nous n'aurions pas l'Euro, et sans l'Euro aujourd'hui, on serait sans doute dans une situation extrêmement défavorable, si vous avez été élu ou votre candidate à l'étude à cinq ans serait sortie de l'Euro alors ah ça aurait été la catastrophe et demander à nos amis britanniques, si aujourd'hui ils se sentent bien mieux, nous n'aurions pas de plan de relance aujourd'hui européen qui a permis à l'Europe de répondre de manière extrêmement forte à la crise sanitaire, nous n'aurions pas acheter des vaccins, ensemble, nous aurons sans doute des pays aujourd'hui en Europe qui serait bien moins vaccinés que le nôtre. Résonance en cela peut-être avec certains pays, dont vous êtes plus proche et puis enfin la défense et la réaction face à la crise ukrainienne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, moi je suis extrêmement fier que la France aujourd'hui avec des enjeux souveraineté importants, ce qui s'inscrit dans un cadre européen de coopération pour faire de l'Europe une une une zone, effectivement qui va être un exemple pour le monde, en terme de développement économique, financier, environnemental et social alors ensuite quand vous rentrez dans le détail, vous parlez de liberté et d'autonomie et de protection notre triptyque nous y répondons, peut-être avec des oeufs, des objectifs et des outils un peu différentes des vôtres, mais la liberté, nous les défendons, peut-être même un peu plus que. Vous si vous étiez au pouvoir, l'autonomie, c'est ce que nous renforçons via toutes les stratégies que j'essaie de vous présenter ce soir, et enfin la protection ne nous dites pas que non pas protégé les Français, ça fait 5 ans que nous le faisons de manière extrêmement forte sur les dit tout à l'heure sur l'inflation, je pense que notre bilan en terme de gestion de la crise sanitaire, on n'en a pas à rougir, franchement, je pense que la France aujourd'hui, fait plutôt partie des nations qui ont plutôt bien géré les crises successives et heureusement que le président, il était à la manoeuvre, plutôt que d'autres, merci. Monsieur le. Président, monsieur le Ministre, chers collègues, souveraineté économique en France et même en Europe, c'est un vaste débat politique qui concerne des modèles économiques et sociaux que les rapporteurs sont ont ouvert et je veux saluer l'excellence de leur 5 plans de reconstruction. va nous nous y engager, nous devons poser les un jeu, un jeu d'indépendance et de liberté, de faire le choix, des choix, un jeu d'emploi et de formation à un jeu de savoir-faire et d'expertise, un jeu de revalorisation des métiers à suite le constat sans appel, si l'on se met des oeillères s'attarde au contexte sanitaire et géopolitique de serre des de ces derniers mois avec le drame de la guerre en Ukraine ces 2 événements ont marqué nos vies chamboulées le confort de nos sociétés, mais non, ils ne sont pas à l'origine de tous les maux, aujourd'hui, qu'il s'agisse de la hausse des prix de la crise de l'énergie, de l'absence d'un produit dans un magasin ou de silence radio, d'une administration, c'est soit la faute au Covid soit la guerre, en Ukraine, les Français, hein, plaisante même conscient d'être berné par des décideurs qui n'assument pas les erreurs du passé, comme elle dit que très bien ce rapport, l'absence de masques n'a fait que révéler une absence de stratégie plus ancienne aux cru une crise et n'est anticipé, et la France a vu son indépendance énergétique industrielle, agricole s'étioler au fil des décennies, pas assez de culture de prospective, pas d'analyse des risques, la France s'était engagée d'un d'une désindustrialisation et dans l'appel des sirènes produire au moindre coût et délocalisée au sein de cet hémicycle, nous relayons pour débattre alerter car l'objet : l'objet n'est pas de jeter la Pierre, mais d'apporter la Pierre à l'édifice pour co-construire je m'attacherai à décliner 5 domaines notre politique commerciale tout d'abord, il va falloir que l'Union européenne montre sa détermination face à certains à certains pays que l'on dit émergea mais qui vont nous submerger comment en adoptant des règles qui protège les entreprises du de l'Union pour l'heure, notre compétitivité, d'ailleurs, ça a été dit quid du et de son débat ou non au Sénat et les autres accords à venir l'approvisionnement ensuite pour l'agriculture, la France est fortement dépendante des protéines végétales car le choix a été déporté, plutôt que de produire, ça me prévoir aucunement les conséquences idem concernant les substances chimiques et les métaux critiques aujourd'hui nous le payons au prix fort, pourquoi Sarko dans des postures politiciennes plutôt que à partir de Costa évident repenser nos modèles par filière, troisièmement la protection nos, nos entreprises, nous détenons une grande richesse, un expertise scientifique médicale dans l'innovation, mais là ce de paperasserie de blocage de lenteurs dans les procédures franco-française, beaucoup d'entreprises font le choix de s'expatrier des cerveaux des savoir-faire qui disparaissent et cela n'est pas admissible il faut plus de simplification administrative, j'avais fait l'expérience de réunir les chefs d'entreprise héraultais d'univers différents hôtellerie de luxe, services médicaux horticulture, énergies renouvelables, entreprises de l'agroalimentaire, nous avions passé à la loupe, des mesures de simplification résultat ces décideurs ont pointé du doigt les vrais problèmes et les vrais besoins de simplification non identifiés, n'ayons pas peur d'ouvrir de de grands chantiers, même si cela bouscule les institutions et les administrations, n'oublions pas que nous sommes au service de l'intérêt général et oublions les effets d'annonce de baisse soyons enfin performant pour cela, changeons de méthode, sortant de leur bureau, les sachant qu'ils pensaient des stratégies dans l'incident je ne changera pas rien à leurs fins de mois qu'ils aillent dans les champs là les entreprises et les laboratoires pour mieux comprendre moi. Pour l'énergie, l'absence de prospective et nous avons voté 40 % d'énergie fossile à moins pour 2030, mais en donnant, quels moyens quelle feuille de route, le résultat aujourd'hui c'est qu'un total panique nous réouvre ont des centrales à charbon nous rappelons des salariés si la licencié, quelle image pour les citoyens et que dire de la moitié des réacteurs nucléaires fermer certes et des accidents de Tchernobyl et de Fukushima certes le choix politique de l'Allemagne de sortir du nucléaire nous ont rendus frileux mais comment abandonner une solution avoir d'avoir totalement abouti les autres concernant le numérique, ça a été dit, il faut absolument une prise en compte et une prise de conscience européenne pour ne plus dépendre des gaffes, hein, ah, en fait, les compétences et métiers de demain un perdant notre Leadership nous perdons aussi nos métiers, nos savoir-faire, la formation, mais aussi l'orientation scolaire sont essentiels, le problème de la souveraineté et transversale, tous les ministères doivent être s'y associer, vous l'aurez compris ce rapport ouvrent des perspectives pour qu'il ne soit pas un rapport de plus, nous attendons une détermination de ce gouvernement, a étudié et suivre ses propositions, partageant les Costa définition les âges réunissant les parties prenantes à la gestion avec les moyens réels, vous l'avez déjà fait avec les états généraux de l'alimentation et de la justice, mais Bercy ne doit pas décider ne doit pas décider c'est aux politiques de gouverner en fonction des âges, sinon la France perdra le peu de souveraineté qui, du reste, et ce n'est pas ce que collectivement nous voulons. Merci monsieur le président, monsieur. Le sénateur Cabanel. Bon, quand je me compare, je me console quand même je pense qu'on a tous une aptitude à se battre la coulpe collective qui est à notre honneur mais oui pendant 25 ans, la France et d'industrialiser oui on a eu une difficulté à anticiper la plus grave crise sanitaire depuis 100 ans. Quand on compare la réaction de la France à cette crise sanitaire et plus largement d'ailleurs celle de l'Europe, je pense qu'on peut être plutôt assez fier du résultat, ça veut pas dire qu'il ne faut pas tirer des leçons, et c'est d'ailleurs l'objectif de ce rapport et c'est ce qui m'a plu, ce rapport, ils se projettent essentiellement vers l'avenir et moi je vous engage à le faire maintenant battre notre coulpe c'est bien regretter les 25 ans, désindustrialisation, c'est bien aussi, il faut qu'ensemble, on travaille pour réindustrialiser la France, et vous avez raison, partout dans les territoires, moi au moins une fois par semaine, je suis dans un territoire pour visiter des usines, des entreprises, certaines qui vont très bien et qui sont là aujourd'hui dans une logique de développement extrêmement porteuse et ça, il faut en être fier, et d'autre, monsieur le sénateur guerre n'a mentionné une ou deux tout-à-l'heure et Duralex que j'ai visité, qui font face à des situations difficiles et c'est vraiment en tenant les 2 bouts, accompagné des entreprises en 3D en transition dans les secteurs difficiles et continuer à accompagner les secteurs d'avenir qu'on va réussir à réindustrialiser la France, vous parliez de la simplification administrative, ce sera un de mes combats également, je pense qu'on peut faire des choses déjà à droit constant, mais on s'interroge avec Bruno Lemaire et on aura sans doute l'occasion d'échanger avec vous sur ce sujet, sur l'opportunité ou pas de passer par la loi, pour simplifier, de manière drastique les, les, les installations industrielles, mais je suis sûr que ça soulèvera sans doute beaucoup de débats, sur ces bancs et sur les autres, mais en attendant on souhaite accélérer au cas par cas, moi j'ai demandé à ce qu'on cartographie le foncier de manière extrêmement fine partout en France pour qu'on puisse proposer à des investisseurs nationaux ou internationaux du foncier catégorisé conséquent correspondant à leurs besoins, on travaille avec les régions, les départements et les communautés de communes pour rendre ce foncier disponible, vous savez on a identifié un certain nombre de sites industriels clés en main qui sont aujourd'hui disponible, bref, nous sommes au travail pour simplifier les installations industrielles et je le répète, ce sera partout et ce sera pour tous et pour toutes, merci. ayant davantage de de la culture de prospective pour effectivement se positionner les voir un petit peu plus loin, il a fallu qu'on connaisse tous ces événements pour savoir combien la France était dépendante donc aujourd'hui, il faut travailler, bien sûr, j'ai insisté sur la simplification, ça me paraît mais aussi au fil du temps, essayons de voir les 2 évaluer aussi les politiques que nous mettons en place pour pouvoir corriger éventuellement les erreurs que nous avons fait pour ne plus connaître la situation dans laquelle nous sommes. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Serge Babary pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame, monsieur, rapporteur, mes chers collègues, le constat dressé par le rapporteur et très alarmant ce travail approfondi confirme malheureusement les inquiétudes que nous exprimons au sein de la commission des affaires économiques depuis maintenant de nombreuses années la crise sanitaire, a mis en lumière ce que nous redoutions, notre économie et de plus en plus dépendante et vulnérable je me bornerai à aborder la question de la souveraineté financière en mettant l'accent sur 3 éléments : premièrement, il faut renforcer le contrôle de l'investissement étranger dans les secteurs stratégiques, ça a été évoqué la loi pacte a posé les jalons d'une politique de contrôle, nous devons aller plus loin pérenniser l'abaissement temporaire du seuil de détention, déclenchant le contrôle à 10 % des droits de vote et élargir les secteurs contrôlés abaissement de seuils qui ne doit pas être réservé aux seules sociétés françaises cotées nos PME doivent bénéficier du même degré de protection que nos sociétés cotées, il importe également d'être vigilant sur la question des fonds de pension pendant la crise sanitaire, un tiers des entreprises de taille intermédiaire, les outils ont été approchés par des fonds de pension anglo-saxon qui supposer qu'elles avaient des difficultés et proposer une aide financière avec la délégation d'entreprise, nous voulons d'auditionner le représentant du métier, le mouvement des ETI le chiffre évoqué désormais de 40 c'est donc plus de 2000 entreprises sur nos 5500 ETI qui ont été approché, cela nous impose d'être extrêmement vigilants pour nous prémunir contre ce type de prédation, nous devons renforcer les possibilités d'intervention de fonds souverains nationaux, deuxièmement, il faut évidemment renforcer la commande publique et soutenir les entreprises innovantes ainsi que les Start-Up mais aussi faciliter l'accès de au PMU aux appels d'offres afin que les attributions n'aille pas toujours au grand groupes parfois étrangers la commande publique de s'ouvrir aux PME, cela ne pourra se faire sans l'adoption d'un Small Business act européen a été évoquée par le président Morales Desailly, troisièmement, il est impératif de mettre en place les conditions du maintien des ETI dans nos territoires de chiffres 50 % des ETI sont des entreprises familiales 25 % des chefs d'entreprise ont plus de 60 ans, il est urgent de moderniser la transmission des entreprises pour lutter contre le rachat par des investisseurs étrangers dans une pure logique de captation de brevets et de savoir-faire, sans considération de la pérennité de l'entreprise elle-même, ou de l'emploi dans le territoire, je souscris évidemment pleinement à l'objectif du gouvernement de faire émerger 500 ETI pendant ce nouveau quinquennat mais la question de la transmission et donc du maintien des ETI existantes reste entière sur ces 3 éléments de défense de la souveraineté financière le contrôle de l'investissement étranger, le renforcement de la commande publique et le maintien de nos ETI, il faut maintenant des réformes structurantes, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, merci. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, barbarie, je vais vous corriger sur une chose : vous trouvez ce rapport alarmant, moi je le trouve extrêmement motivant, je souhaite véritablement qu'ensemble, en partant de constats qui sont juste qui sont sévères mais qui sont, finalement, le dessin de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, on se mette d'accord pour aller de l'avant, la France a des forces, la France a des atouts, on a je suis désolée, mis en place un certain nombre de choses depuis 5 ans qu'ils nous ont permis d'inverser un certain nombre de tendance qui jusqu'alors apparaissait inéluctable, moi j'ai commencé à travailler au ministère de l'Économie et des finances, il y a 30 ans, politique industrielle, c'était un gros mot, à l'époque, il y en avait que pour la politique macro-économique, la politique monétaire, la mise en place de l'Euro, je le répète, excellent choix stratégiques et historiques. Mais qui n'a pas empêché la désindustrialisation ça changé aujourd'hui, nous sommes prêts, les investissements étrangers en France, vous l'avez dit, nous avons renforcé la législation nous les contrats longs, n'oublions pas pour autant que l'attractivité de la France fait partie de ces atouts aujourd'hui, vous parlez des fonds de pension anglo-saxon, moi je vois presque chaque semaine des grands investisseurs étrangers qui sont des investisseurs opérationnel des grandes entreprises pharmaceutiques, des grandes entreprises chimiques des grandes entreprises industrielles américaines asiatiques qui souhaitent venir investir en France parce que notre pays est très attractif, il faut le garder à l'esprit ça et donc quand on. La fin notre politique de protection des intérêts stratégiques, il faut quand même garder cela à l'esprit, moi je pense que ce qu'on a fait dans la voie pas qu'est un bon équilibre, je l'ai dit tout à l'heure, ça a déjà commencé à donner des résultats, j'entends que l'histoire du 10 pour reste à préciser pour l'instant ce seuil de 10 % est valable jusqu'à la fin de l'année, on devra évaluer si on doit le pérenniser ou pas et ça fera partie, sans doute des discussions qu'on aura ici du côté du manque d'investisseurs institutionnels, vous avez raison, moi j'ai été numéro 2 d'une grande caisse de retraite québécoise pendant 10 ans, qui était le plus gros investisseur dans les entreprises québécoises et qui permettaient de développer des PME et des ETI on en manque encore cruellement d'investisseurs publics de long terme, en France, on a créé la BPI qui est quand même un acteur reconnu, on a créé aussi, sous l'égide du président de la République, une initiative qui ont fait que les assureurs français se sont impliqués, je pense que c'est le fond, qu'on appelle le fond Tibi qui à hauteur de 6 milliards d'euros investis aujourd'hui dans des entreprises de taille modeste en France, avec vocation les accompagner, on doit aller plus loin, je ne pense pas qu'on ouvrira le sujet des fonds de pension en France, je dis ça pour réveiller Monsieur le Sénateur gain qui à mon avis il serait heureux de l'entendre, mais évidemment, nous devons trouver du capital de long terme n'est pas disponible sous la forme de retraite, nous devons trouver d'autres moyens, les assureurs feront sans doute partie des candidats merci. Merci, Monsieur le Ministre Monsieur bah Marie une réplique. Monsieur le Ministre, merci de de de vos propos, quand on sonne l'alarme, c'est évidemment un constat d'un certain nombre d'inquiétudes, mais c'est aussi parce que on souhaite par ambition pour notre pays, avec vous, se projeter dans l'avenir, on n'est pas tourner simplement dans le constat de des difficultés passées cette alarme, elle est aussi ce que nous entendons sur le terrain, dans notre travail de de d'élus dans dans nos territoires et donc on fait le par le porte-parole, les porte-parole plutôt des PME et ETI qui sont un petit peu laissé de côté leurs sentiments, alors que, on a des chefs d'entreprise très entreprenant plein de, de volonté de développement leur sentiment, c'est quand même que les facilités sont plutôt pour les grandes entreprises et d'ailleurs, le lien entre les grandes entreprises et les plus petites, si on se compare avec des pays voisins comme l'Allemagne ou l'Italie, où nous avons fait le déplacement pour voir comment fonctionnait le système et le succès à l'exportation, il travaille en meute, c'est-à-dire que la grande entreprise entraîne dans son sillage les PME et ETI, c'est ça que nous souhaitons, et c'est ça le le sens de notre à la mer. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Sébastien Pla pour quatre minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission, madame, monsieur, là, le rapporteur, mes chers collègues. Je le 3ème pilier de notre économie, l'agriculture française avec 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires reste en valeur la première puissance agricole de l'Union européenne, devant l'Allemagne et l'Italie, mais derrière cette comparaison flatteuse, se cache une réalité bien plus inquiétante, l'excédent de notre balance agricole est assise essentiellement sur la production Viti Viti vinicole, la moitié des produits qui sont dans notre assiette sont emportées et la France reste par ailleurs dépendantes à 45 % de l'étranger pour les protéines végétales depuis plus de 20 ans, la production agricole française recule, nous avons perdu 25 pour 100 des parts de marché et les agriculteurs déserter les campagnes 10000 exploitations agricoles disparaissent tous les ans il faudrait chaque année 7000 nouveaux agriculteurs pour compenser les départs à la retraite, le métier n'attire plus, cette crise de vocation est associé à la question de la fracture territoriale aux difficultés de la vie hein jaune rural face au retrait des services publics, aux difficultés d'accès aux soins, aux transports et au numérique, mais elle est aussi et surtout lié à la faiblesse des revenus de celles et ceux qui cultivent la terre, les aides PAC deviennent pour bien des fermes, la majeure partie du revenu la PAC est complètement décorrélé de la création de valeur ajoutée et ne parvient pas à relier les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation, dans un contexte géopolitique mondial tendu, nous devrions redoubler de vigilance pour garantir la transparence sur l'origine et la qualité des produits distribués sur le marché, ainsi que notre sécurité alimentaire, de nombreux outils pourrait être activé, comme l'instauration des clauses miroirs dans les accords de libre-échange ou encore une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, car manifestement aujourd'hui il est demandé aux producteurs français de réussir un exploit, celui d'adapter des pratiques toujours plus durable mais coûteuse tout en rivalisant avec des systèmes d'élevage intensif, notamment venant du continent américain, la France qui a fait le choix, par exemple pour l'élevage d'un élevage durable et familial ne peut continuer d'accepter une mise en concurrence de ces exploitations avec des fermes usines américaines de 60000 bovins engraissés aux antibiotiques que le risque de retrouver dans nos assiettes, grâce à ce super d'accord que le site si nous voulons assurer la sécurité alimentaire des Français, tout a maintenant notre rang de 1er producteur agricole de l'Union européenne de nouvelles politiques alimentaires et agricoles s'impose, il faut qu'elle soit en phase avec les enjeux du moment, sans obérer les stratégies farm to forte de l'Europe, nous devons de faciliter les conditions de travail de nos exploitants en garantissant leurs revenus en accompagnant la transition agroécologique en pérennisant des dispositifs, notamment le TO-DE, pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre, nous devons relocaliser l'ensemble de la chaîne de production, à commencer par les train jusqu'à la transformation et l'emballage, mais aussi hein reterritorialisation la consommation, il faut aussi en finir avec la surtransposition des règles et des normes par rapport aux autres pays européens, car à chaque nouvelle contrainte imposée aux seuls producteurs français se succèdent une vague d'importation de produits étrangers, vous savez comme moi que la France exporte des animaux entiers et des morceaux découpés, vous savez comme moi que la France exporte des pommes de terre et emportée Chips vous savez comme moi que la France exporte du blé et un porte de la farine et des pâtes, cela n'est plus logique et encore moins acceptable, donc une politique de patriotisme alimentaire doit être véritablement assumer pour répondre au double enjeu de souveraineté alimentaire et de lutte contre le changement climatique, mais attention à à trop nous focaliser sur le soutien à la production, nous oublions de renforcer nos capacités de transformation indispensable à la conquête de nouveaux débouchés, gage de création de valeur et de compétitivité, le risque est une incitation à s'approvisionner ailleurs, voir une désindustrialisation agroalimentaire accélérer si l'agriculture elle n'est pas délocalisable l'industrie les avec d'autant de conséquences pour notre souveraineté alimentaire, enfin, Monsieur le Ministre, n'oubliez pas l'importance d'être fort sur le marché domestique pour être compétitif à l'extérieur et que les réponses politiques devront aussi été de n'être qu'agricole pour devenir agricole, agroalimentaire et alimentaire, le secteur agricole, un fleuron de notre économie et de notre souveraineté est actuellement en grand danger. Merci, merci, cher collègue, la parole à Monsieur le Ministre. Merci, merci Monsieur le Président merci monsieur le sénateur plat alors vous êtes sortis un peu de ma zone d'excellence puisque vous avez essentiellement consacré votre intervention, l'agriculture, que j'ai suivi de près, quand je présidais la commission d'affaires économiques

c'est plus de 600 millions d'euros d'investissement qui ont d'ores et déjà été consacré et dépensés pour améliorer notre souveraineté alimentaire, on a aujourd'hui 5 % de moins, c'est pas grand chose mais c'est quand même ça de dépendance vis-à-vis des protéines végétales, on a relocaliser un certain nombre d'intrants critique et on va continuer à le faire dans le cadre de France 2030 ces deux 3 milliards d'euros qui sont destinés à la relocalisation des tourteaux, des acides aminés, des engrais, et est-ce qu'il faut fermer les frontières françaises à l'agriculture française et ce qu'il faut essentiellement rester dans une logique d'auto-suffisante, je ne crois pas, je ne suis pas sûr qu'il faille fabriquer toutes les pâtes alimentaires françaises qu'on mange en France en France, parce que moi je suis persuadé que l'agriculture française peut reprendre des couleurs à l'international, aujourd'hui, vous l'avez dit certains, d'autres l'ont dit avec vous, la balance commerciale agricole s'est fortement détériorée depuis des décennies, ce n'est pas une fatalité, nous devons investir davantage dans l'agriculture, la rendre plus efficace la rendant peut-être aussi peut être peut être mieux connu parce que vous l'avez dit le modèle agricole français qui est souvent basé sur la qualité, sur des exploitations de taille réduite était insuffisamment marqué je dirais à l'international, vous allez dans un supermarché à peu près partout dans le monde, vous allez trouver un rayon italien. Vous allez dans un supermarché à peu près dans le monde, vous allez parfois trouver du bris du Bordeaux ou du Bourgogne et je ne veux pas faire de jaloux malheureusement je ai cité fromages et de vins mais la la la nourriture française l'excellence française, je pense qu'on doit faire mieux pour la vendre en tant que telle, la marque France de l'agroalimentaire, moi je suis persuadé qu'elle doit pouvoir faire mieux et j'en ai déjà parlé avec mes collègues Faynot et Best et je pense qu'on va y travailler et donc, si on veut pouvoir exporter la marque France il va aussi pouvoir parfois hein porter la marque Italie ou la marque espagnole, peut être qu'on apportera toujours des pâtes italiennes mais j'espère qu'on exportera de plus en plus de nourriture française merci. allez-y chers collègues. c'est tellement bien que, aujourd'hui, ça fonctionne pas tout à fait correctement, nous avons de moins en moins d'agriculteurs, nous continuons à faire des exploitations sur tous les niveaux, et je le voulais dit en entrée, la balance l'excédent balance commerciale et repose sur la viticulture, essentiellement, qui ne sont pas aujourd'hui des produits de nourriture et agroalimentaires au sens nécessaire pour la vie humaine, la question qui est posée, c'est la souveraineté alimentaire donc quid des produits des céréales de de l'élevage et de l'ensemble des productions, des tomates, tous les produits du maraîchage comment relocalisé sur le territoire français pour éviter à la fois n'aime pas carbone qui est catastrophique pour la planète et ensuite de dépendre de marché qui aujourd'hui sont à l'extérieur et très sensible, voilà. Merci, la parole est maintenant à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour 4 minutes. 4 minutes. Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, parmi les 5 axes déterminant pour la souveraineté de notre pays, nos 3 collègues dont je salue le travail ont bien évidemment développer le sujet numérique, je voudrais revenir sur ce cet enjeu incontournable pour nos sociétés d'information on nous projetons dans l'avenir, Monsieur le Ministre et en y ajoutant la dimension spatiale en effet alors que dans de nombreux champs du numérique, notamment les donner notre souveraineté française et européenne est compromise par la domination des Gafam, les Big Five et autres BATX asiatique en matière de réseau et de spatial, les cartes ne sont pas encore joué et la conquête d'une souveraineté européenne reste possible, comme l'a bien compris notre commissaire européen Thierry Breton très investi sur ce sujet, les récents travaux de nos commissions Affaires économiques et affaires européennes nous éclaire tout particulièrement sur les enjeux de souveraineté liés au projet de constellation européenne de satellites, la proposition de résolution européenne du Sénat met en évidence tout l'intérêt d'assurer une connectivité sécurisée indépendante pour les usages gouvernementaux, notamment militaires, mais également pour les usages commerciaux, la chirurgie à distance les véhicules autonomes, le guidage de précision des bateaux, des avions ou, plus pratiquement la couverture des zones blanches des territoires ultramarins le Sénat préconise une approche stricte de la préférence européenne, autrement dit les satellites de la constellation européenne devront être déployés par des lanceurs européens depuis des bases de lancement situé sur le territoire de l'Union européenne, il s'agit là d'un enjeu primordial de maîtrise de nos télécommunications mais aussi un levier pour bouster technologiquement et financièrement nos industries, affirmé la préférence européenne en matière d'infrastructures spatiales, c'est soutenir le développement et l'innovation des industries spatiales française et européenne, les acteurs pivot historiquement établis, mais aussi faire émerger des Start-Up du New Space est à même d'apporter des solutions sécurisées aux entreprises comme aux particuliers, au service public sait enfin soutenir le déploiement de nouvelles technologies numériques émergentes comme, par exemple, ça a été évoqué le Cantique, bref la constellation européenne de satellites constitue une brique essentielle dans le modèle économique européen du XXIe siècle, bien au-delà du spatial, Monsieur le Ministre : quelle place demain pour la France et l'Europe à la table des relations internationales si, contrairement aux autres grandes puissances, elle ne dispose pas d'une constellation de satellites autonome, comment pourrions-nous concevoir le déploiement d'un le déploiement d'infrastructures spatiales gouvernementales par des lanceurs américains ou des acteurs extra-européens mais cette préférence européenne stratégique ne se fera pas sans engagement réciproque de la part des entreprises et de l'industrie spatiale européenne afin qu'elles assurent la cadence et la fluidité des lancements européens mais aussi des opérateurs d'infrastructures terrestres européens qui devront être en capacité d'accueillir ces nouveaux flux de connectivité dans des délais serrés car, Monsieur le Ministre, si l'Europe veut accueillir ses acquérir cette souveraineté en matière de tes que les communications, elle doit aujourd'hui faire vite, déjà 2700 satellites Starlink sont en orbite de pour le la constellation Gwenwed et la consolation Cooper d'Amazon est en phase de lancement par Ariane Espace, monsieur le ministre, la préférence européenne et même la localisation dont nous parle le long beaucoup constitue-t-elle, selon vous, un véritable rempart notamment face au regard du droit extérieur extraterritoriaux notamment du droit européen évoqué aussi par nos collègues dans ce rapport qui fait toujours planer des des menaces de contrôle et de sanction sur nos fleurons technologiques du simple fait de l'usage du dollar dans les transactions, je remercie vraiment je salue le travail de nos collègues qui pointe avec réalisme nos faiblesses à compenser tout autant que nos atouts à valoriser, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Loisier elle est là, le moment que je craignais est arrivé, je n'ai pas de réponse à vos questions en tout cas pas de réponse à mon goût satisfaisante, on me dit, évidemment qu'il y a plusieurs projets de constellations qui existe en Europe, qui vont être lancés hein par Thales et Télésat pour 3 milliards d'euros, un autre qui vise à créer une constellation de satellites et 5 G et que la commission a annoncé en mars dernier un projet de constellation, j'ai bien conscience que cette réponse est assez insuffisante, donc je m'engage à vous aurez une réponse plus circonstanciée par écrit, si vous m'y autorisez dans les jours qui viennent. Allez-y, chers collègues. vous enquérir de ce rapport parce qu'effectivement je pense que tout ce que nous évoquons aujourd'hui c'est largement conditionnée à notre véritable souveraineté sur nos télécommunications et le spatial et la voie royale demain pour les télécommunications, merci. Merci, cher collègue, et la parole est maintenant au président Jean-François Rapin pour. Cinq minutes, ce sera le dernier intervenant. monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, madame et monsieur le rapporteur, il est effectivement urgent pour notre pays de reconquérir sa souveraineté au plan économique, nous savons gré la commission des affaires économiques et sa présidente et au rapporteur d'avoir tiré la sonnette d'alarme, je ne reviendrai pas sur leur excellent rapport, je veux simplement rappeler que la France a accepté de partager en partie sa souveraineté avec les autres États membres de l'Union européenne et qu'à ce titre, la reconquête de sa souveraineté se joue largement à l'échelon européen, il aura fallu la crise sanitaire et le conflit et le conflit ukrainien pour prendre la pleine mesure des dépendances stratégiques de l'Union européenne et des fragilités et menace qu'elle constitue pour ses citoyens et ses entreprises

européenne en matière de défense mais aussi de santé d'alimentation d'énergie de matières premières critiques de numérique de technologies fondamentales et Anne Catherine la rappeler 2 spatial, c'est un chantier au long cours, mais il est heureux que l'Union européenne, on est fini avec la naïveté, enfin, car ce n'est qu'à cette échelle que nous pouvons espérer construire une souveraineté durable, l'Union est aujourd'hui entrée dans le réarmement de ces politiques avec tous les outils dont elle dispose, concurrence, financement politique commerciale des projets importants d'intérêt européen commun ont été lancés, qui dérogent aux règles en matière d'aides d'État pour promouvoir l'innovation dans plusieurs domaines industriels stratégiques batterie semi-conducteurs Claude hydrogène autant de Piak, auquel l'industrie française participe le prochain Chips acte doit aussi permettre à l'Europe de redevenir leader mondial des semi-conducteurs et la présidente de la Commission européenne promet un nouveau fonds européen pour la souveraineté qui permettra de financer d'autres projets industriels stratégiques. Pour sécuriser nos approvisionnements en matières premières critiques un plan européen vient aussi d'être annoncée de textes européens majeurs pour réguler les marchés, ça été rappelé et services numériques le DMA et le DSA ont été récemment adopté, il constitue également des outils importants de reconquête de notre souveraineté en en ce domaine, saluons enfin en matière spatiale, la création prochaine d'une constellation de connectivité sécurisée européenne, monsieur le Ministre, en lisant le rapport, vous serez au fait de l'actualité, pleinement, en outre, pour protéger le le marché intérieur, de la concurrence déloyale, un règlement sera bientôt adoptée qui mettra fin aux subventions étrangères faussant la concurrence pour sauvegarder nos industries stratégiques du point de vue de l'ordre public et de la sécurité, un cadre commun a aussi été mis en place permettant de filtrer les investissements Directs étrangers dans l'Union, la commission des Affaires européennes, soutient vigoureusement toutes ces initiatives et prend soin de les orienter, elle plaide aussi pour aller plus loin, d'abord en matière énergétique, l'envolée des prix de l'énergie nous menace d'une nouvelle vague de désindustrialisation et risque de briser le sursaut provoqué par la pandémie en Allemagne et maintenant en France, des usines ralentissent étranglés par leur facture énergétique, ce qui freine la relocalisation des chaînes de valeur tout récemment engagé tout en soutenant une réforme du marché européen de l'énergie, nous appelons l'Union européenne à reconnaître, sans attendre le nucléaire comme une pièce maîtresse de la transition et de la souveraineté énergétique européenne car il s'agit d'investissement de très long terme, nous subissons aujourd'hui le choix de nos voisins, de produire leur électricité à partir du gaz, je crois qu'il mettent à mal aussi bien nos objectifs climatiques que notre compétitivité et notre indépendance énergétique degrés qui a fait le gouvernement sur la question nucléaire je relisais tout à l'heure, les minutes de certaines commissions d'ailleurs que vous présidiez où la question du nucléaire n'était pas aussi clair qu'elle est aujourd'hui. Ensuite en matière agricole, nous ne cessons de le répéter, ne sacrifions pas notre souveraineté alimentaire sur l'autel de la transition écologique, nous ne pouvons pas nous ranger à une vision décroissante de notre agriculture et limiter notre stratégie agricole a encouragé la montée en gamme de nos filières, au risque de devoir accroître nos importations, enfin en matière bancaire et financière nous rappelons la nécessité de consolider ce qui est la colonne vertébrale de notre souveraineté économique, il s'agit d'abord d'achever le dernier pilier de l'union bancaire pour améliorer la résilience des banques de la zone Euro, ce qui passe par un système européen de garantie de dépôts, il s'agit aussi de relancer l'Union des marchés de capitaux pour mettre fin à la fragmentation des marchés financiers européens, il importe enfin de consolider le rôle international de l'Euro, vecteur de souveraineté sur ces différents sujets, nous portons haut et fort la voix du Sénat à Bruxelles au service d'une souveraineté retrouvée, Monsieur le Ministre, pouvons-nous aussi compter sur la détermination du gouvernement pour porter ses priorités, je n'en doute pas, à vous écouter ce soir.

monsieur le président merci au président hein pour pour son intervention à laquelle je souscris à 98,5 % je pense, et pour le reste, j'aurai la réponse bientôt évidemment nous avons un agenda européen extrêmement ambitieux évidemment tout ce dont nous parlons ce soir doit s'inscrire, je pense que la plupart d'entre vous en êtes convaincu dans un cadre européen extrêmement, extrêmement ambitieux, peut-être pour conclure, de mon point de vue, ce débat, monsieur le président, madame la présidente, Prima madame la rapporteure, quinquer et monsieur le rapporteur Montaugé merci encore pour pour votre travail, quand on parle d'industrie française c'est qu'on porte tous le même maillot, je l'ai dit dans cet hémicycle, ou dans d'autres, sur les bancs de gauche ou sur les bancs de droite dans ma position dans la vôtre. Certes, certains élus d'un extrême, ou d'un autre n'aime pas beaucoup l'entreprise, il n'aime pas beaucoup l'industrie soit parce qu'ils ne la connaissent pas, soit parce que pire, ils doivent en partie leur succès au déclin de l'industrie depuis des décennies, mais ici au Sénat après avoir entendu vos différentes prises de parole, je crois pouvoir dire que presque tout le monde ici M. l'industrie française et pour l'essentiel, nous sommes alignés sur nos objectifs, j'ai partagé plusieurs des constats formulés dans votre rapport, je ne vais pas m'y attarder mais sur les recommandations, la plupart, je le répète, sont déjà elle aussi mise en oeuvre où figurent dans ma feuille de route, je vais être ici extrêmement clair, en revanche, la protection oui le protectionnisme non l'industrie française pour être forte, elle doit être solide sur ses bases, mais elle doit être aussi capable de conquérir des marchés dans une logique de réciprocité loyal, un certain nombre de dans d'entre vous ont insisté sur ce loyal et je pense qu'il est important, cette industrie française, elle doit être aussi capable d'attirer des investisseurs internationaux tous France est une vraie réussite, nous allons accélérer nous sera utile, je tiens à dire par le panorama qui l'établit et je pense qu'il dresse aussi une feuille de route de nos collaborations à venir, on l'a dit, notamment sur des sujets extrêmement concrets comme celui de la simplification des installations industrielles, j'aimerais pour terminer affirmé mon engagement très fort à agir sur 2 points : le 1er, un certain nombre de d'entre vous l'ont mentionné et il est régulièrement évoquée dans le cadre de ce rapport, c'est la mobilisation de la commande publique, nous avons voté ensemble, j'étais à l'époque député donc je peux utiliser ce nous des dispositions très concrètes dans la loi, pacte dans la loi dite ASAP ou dans la loi climat résilience, il faut aujourd'hui les appliquer trop souvent les acheteurs publics n'osent pas les utiliser, nous devons les rassurer sur le fait que oui nous devons acheter durable, nous devons acheter innovants et oui, nous pouvons acheter local et en circuit court. Durable innovant local en circuit court, c'est peut-être pas forcément systématiquement acheter français mais ça commence à y ressembler. J'ai déjà rencontré mobiliser la direction des achats de l'État, l'Union des groupements d'achats publics et des acheteurs publics nous allons former davantage faire du sourcing promouvoir nos Start-Up et PME et faciliter les échanges en amont des procédures. Sur la formation, je serais plus bref, mais un certain nombre d'entre vous l'ont mentionné nous devons accélérer, c'est un impératif le quinquennat qui s'est achevée il y a quelques mois, a engrangé un certain nombre de succès, on sait, on a jamais eu autant d'apprentis en France, on en a autant qu'en Allemagne, on doit aller plus loin, on doit former des jeunes et des plus jeunes qu'aujourd'hui encore aux métiers de l'industrie, nous devons ensemble donner envie aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de rejoindre l'industrie, je m'y attacherai et j'espère que de ce point de vue-là comme sur d'autres, vous nous y aiderez. évidemment, notre industrie connaît une actualité forte avec la crise de l'énergie qui agit comme un nouveau choc pétrolier, sur ce point, je veux être très clair, l'industrie française ne sera pas la victime collatérale de la guerre en Ukraine, c'est mon rôle de la protéger, c'est mon rôle de l'aider, c'est mon rôle de l'accompagner de la soutenir partout où je le peux, mon cabinet travaillent d'arrache-pied avec les commissaires au Redressement les CRP les femmes CRP dont j'oublie toujours ce que le pays vous dire mais on ne le rappellera les CRP qui dans les régions aident les entreprises à naviguer les dispositifs d'aide encore trop complexes que nous avons simplifié, nous travaillons avec le gouvernement, au niveau national, au niveau européen pour parfaire l'arsenal de protection de l'industrie française. Nous avons signé, ce matin, vous le savez, une charte avec les distributeurs d'énergie, de manière à ce qu'ils informent bien en amont qu'ils offrent systématiques ont des contrats et qu'ils puissent faire jouer la concurrence, appelant notamment à nos PME qui aujourd'hui souffrent de prix de l'énergie trop élevé. Au-delà des mesures ambitieuses que le gouvernement mette en oeuvre pour les entreprises, c'est un fait, les prix de l'énergie ne seront jamais plus aussi bas, c'est la fin d'une disponibilité abondante et sans limite, pardon d'au sein de notre industrie à sa dépendance aux hydrocarbures, il en va aussi du développement d'une industrie de la décarbonation l'industrie de la décarbonation sera le nouveau fer de lance de l'économie française et européenne. Pour terminer, nous avons un cap stratégique nous y affectant les moyens grâce à France relance et grâce à France 2030, nous ne sommes pas naïfs, mais nous sommes offensifs depuis 2017, nous avons créé collectivement avec les chefs d'entreprises industrielles, plus de 50000 emplois neuf c'est un implant vous le dites dans votre rapport, la désastreuse la désindustrialisation pardon a été le résultat d'une cécité collective depuis 30 ans la ré-industrialisation, elle aussi, sera le fruit d'une vision commune, vous y avez toute votre part ici à Paris mais aussi surtout dans nos territoires dans lesquels je me rends, semaine après semaine et où je serai très heureux de vous accompagner, mesdames et messieurs les sénateurs, merci. De votre attention. Merci monsieur le ministre, et pour conclure le débat, la parole est maintenant à Madame Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je suis moins grande que le ministre ça viendra peut-être un jour ou pas, je peux me permettre de de pupitre, monsieur le monsieur le Ministre, mes chers collègues corapporteur et et chers collègues, je vous remercie sincèrement de tous ces échanges et cette prise de parole qui nous ont permis, je crois, de partager, d'approfondir les conclusions de ce rapport avant de conclure : je souhaiterais revenir moi aussi quelques instants sur la question de notre souveraineté énergétique qui appellent de ma part quelques commentaires sur notre politique monsieur le Ministre, il est urgent urgentissime même de définir enfin une véritable stratégie de l'énergie et un cap clair, malgré les belles paroles que j'ai entendu ce soir très optimiste, je ne vois pas la preuve de l'engagement du gouvernement sur cette voie, je regrette par exemple que le gouvernement ait choisi de légiférer en la matière, dans la panique et dans le désordre dans la panique d'abord lorsque le le gouvernement nous a demandé de légiférer dans l'urgence cet été 15 jours d'examen sur une loi sur le pouvoir d'achat pour remettre à plat notre régulation nucléaire notre sécurité d'approvisionnement, clairement, ce n'est pas sérieux dans le désordre, ensuite, oui, Monsieur le Ministre, car il a, il eut fallu examiner la loi de programmation de l'énergie d'abord, pour définir une véritable vision de notre politique énergétique et, ensuite, ensuite seulement travailler aux lois d'exécution de cette stratégie, via les projets de loi d'accélération du nucléaire ou des énergies renouvelables, nous faisons l'inverse au regard de ses impacts la politique énergétique ne s'improvise pas, elle nécessite une une vision des convictions du courage, de la constance et de l'anticipation, or s'agissant par exemple de la relance nucléaire dont nous avons parlé plusieurs fois ce soir tant attendue, elle est encore au milieu du guet des fautes graves ont été commises dans le passé, très bien, mais la reconversion pré-électorale du président n'y a rien changé, les annonces de discours de Belfort sont très insuffisantes, notre commission à évaluer les besoins et monsieur à 14 réacteurs contre 6 annoncé et la nécessité de développer massivement l'hydrogène issus de l'énergie nucléaire n'a pas été clairement annoncée, pour cela nous devons redonner à la filière des moyens financiers, certes, et cela a commencé, mais aussi des moyens humains et une perspective positive positive d'avenir pour nos jeunes, sur les énergies renouvelables, que dire si ce n'est que le Sénat vous pressent d'agir depuis 2020, notre commission a fait adopter 30, solution de simplification dans les domaines de l'hydroélectricité de l'hydrogène du biogaz de l'éolien du photovoltaïque et dans ce rapport, nos travaux se sont penchés sur 2 impensé du renouvelable, l'insuffisance du stockage des énergies renouvelables et notre dépendance minière en bateau, on métaux stratégiques indispensable, c'est aujourd'hui un débat à huis clos, c'est un débat d'experts, je le crois, il faut le partager avec les Français en responsabilité, expliquer à nos coûts citoyen qu'il faut bien sûr recycler, mais qu'il est important aussi de se poser la question de l'extraction notamment du lithium en France, nous allons devenir des gros consommateurs et il nous faut assurer non seulement notre approvisionnement mais aussi prendre nos responsabilités éthiques en étant intransigeant sur les conditions sociales et environnementales de leur extraction, bref, les ménages, comme les entreprises ont besoin d'une énergie disponible abordable décarbonés, c'est une nécessité pour notre vie économique pour notre vie sociale, c'est un impératif au regard de nos engagements climatiques, mes chers collègues, monsieur le ministre, en conclusion, je crois que nos échanges témoignent de 2 choses : d'abord que la prise de conscience et là débattre des vulnérabilités de notre économie n'est plus tabou, c'est regarder en avant et c'est la première étape d'une reconstruction attendu la terre, l'impératif de souveraineté économique est désormais présent dans toutes les têtes, enfin, d'autre part, cette politique de souveraineté n'est pas la la caricature que certains veulent en faire, elle n'est ni repli, ni contrainte ni décroissance ni source de division entre nous, elle est au contraire espoir et elle est faire également européenne européenne cher président, au contraire, sur des sujets comme la souveraineté industrielle comme le numérique comme l'énergie notre assemblée peut et sait transcender les différences politiques ce rapport le démontre, signé à mains, voté à l'unanimité de notre commission, c'est là un objectif partagé de résilience, c'est un projet pour refaire société pour reconstruire sens ensemble le sens de notre nation,

du travail parlementaire, ça n'a pas toujours été le cas, je pense par exemple à la privatisation d'aéroports de Paris dans le cahier des charges, annexé à la loi était une tartufferie à la vente des chantiers de l'Atlantique au débat autour des traités de libre-échange et dans des questions souvent ou encore plus récemment aux discussions sur l'avenir d'EDF Monsieur le Ministre, je réaffirme devant vous au nom de mes collègues de la commission des affaires économiques, que le Sénat est prêt, nous sommes prêts à être force d'engagement, force de propositions pour amorcer la nécessaire reconstruction de notre souveraineté, j'espère que le gouvernement saura se montrer à l'écoute, il se vous permettez, monsieur le Président, je prends une seconde pour remercier l'équipe des administrateurs de la commission des affaires économiques de nous avoir permis de produire un rapport tous ensemble de cette qualité, merci à vous, Sébastien et à votre équipe et merci à mes colistiers merci Monsieur le Ministre, pour ce débat, merci, cher collègue. merci à à tous les participants à ce débat qui ont respecté les les règles et les nouvelles règles de ce débat interactif, mes chers collègues, je vais lever la séance, la prochaine séance aura lieu le jeudi 6 octobre à 10 heures 30 pour les questions orales, la séance est levée.